La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance ? Je n'en vois pas. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, avant d'ouvrir notre séance de questions d'actualité au gouvernement, Je souhaiterais évoquer les événements graves qui ont frappé les consciences au cours des derniers jours. Le meurtre d'une jeune fille de 15 ans poignardée jeudi dernier et les blessures occasionnées à trois de ses camarades dans un lycée à Nantes par un élève de cet établissement. Le meurtre non moins odieux dans le gare d'un jeune fidèle de la mosquée de la Grande Combe poignardée dans un lieu dédié à la prière. Le Sénat exprime toute sa solidarité à la communauté musulmane. L'agression d'arabins à Orléans sortant d'une synagogue devant son jeune fils. Le combat contre l'antisémitisme est une grande cause nationale. Ces faits illustrent l'état de fracturation de notre société. Au nom du Sénat tout entier, j'assure les familles des victimes de notre compassion et de notre solidarité. Ces crimes qui s'ajoutent à ceux commis tous les jours dans un monde toujours plus violent, notamment en raison des conflits de tous ordres qui le parcourent, nous interpellent. Chacun doit doit pouvoir pratiquer, s'il le souhaite, son culte en toute liberté et en toute sécurité. C'est d'ailleurs au fondement de notre République. Notre pays a besoin de retrouver le vivre ensemble qui fait une communauté nationale. Chacun doit y prendre sa part, y assumer ses responsabilités. Il n'y a pas de combat plus noble que celui mené contre le racisme et pour la laïcité. En ces temps difficiles, nous avons aussi accueilli le message de paix légué par le pape François qui fut sa vie durant un homme un homme de dialogue qui n'a cessé d'appeler à la fraternité. Je vous appelle donc mes chers collègues à un moment peut-être de réflexion collective. Face à tout cela, ça me paraît extrêmement important. Oui, réflexion collective et de recueillement. Je vous propose quelques secondes de partager ce moment. Je vous remercie. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et notre site internet. Au nom du Bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges le respect des uns et des autres et bien sûr aussi celui du temps de parole. Je vais donner la parole au président Mathieu Darnot pour le groupe Les Républicains. Premier ministre, vous avez ouvert lundi une séance de concertation sur l'introduction du scrutin proportionnel. Alors, nous savions toujours la concertation. Si nous saluons toujours la concertation, pourquoi cet empressement ? Pourquoi vouloir de ce poison électoral dans une période où les tensions géopolitiques exacerbent les difficultés, où les Français s'inquiètent pour leur On peut vous reconnaître une constance sur le sujet, mais force est de constater que sous la Ve République et bien avant, la proportionnelle n'a généré que de l'instabilité gouvernementale et un régime des partis politiques. Et puis, monsieur le Premier ministre, quelle proportionnelle ? Une proportionnelle intégrale ? Une proportionnelle départementale ? On peut dès lors s'inquiéter pour la représentation des Français qui vivent dans la ruralité, qui vivent en outre-mer. Le vrai sujet, Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas de se concentrer sur l'essentiel, de préparer un budget sans hausse d'impôts, de s'attacher à défendre le pouvoir d'achat des Français, de donner plus de liberté à nos entreprises et de la sécurité pour tous ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président d'Arnaud. La réponse que je vous fais, vous savez à quel point elle est amicale. me... Non, ça démarre très bien. Je viens d'entendre votre charge contre le scrutin proportionnel. dont vous avez dit qu'il était un poison de la démocratie et qu'il était la cause de toute instabilité. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que le scrutin proportionnel, c'est celui par lequel est élu 75% des sénateurs, des membres de cette assemblée, et je n'ai pas le sentiment que ce mode d'élection ait suscité un poison destructeur de la société démocratique, ait suscité l'instabilité. Il suffit de voir ces bancs pour mesurer qu'au contraire, il y a là un facteur de stabilité. Madame, quand vous dites qu'il n'y a rien à voir, il y a tout à voir. Et donc c'est absolument une règle démocratique. Je veux rappeler que tous les pays européens de l'Union Européenne, sans exception, ont ce mode de scrutin. C'est la première chose. Je vais vous dire pourquoi j'ai en effet décidé d'ouvrir des concertations très larges sur ce sujet. Au delà de la constance que vous avez bien voulu reconnaître puisque, en beaucoup de temps dans ma vie politique à militer pour ce changement de nos règles. Pourquoi ? La première de ces règles, c'est parce que la proportionnelle, c'est le scrutin du pluralisme. Et Dieu sait que dans la société que nous vivons, dont le président du Sénat a rappelé à quel point elle était fragmentée, éclatée, opposée, archipélisée, Dieu sait qu'on a besoin d'apaiser la réalité du pluralisme. Deuxièmement, Le scrutin majoritaire, il obéit à une règle simple, il faut être ou tout pour ou tout contre. Et Dieu sait que les problèmes que nous avons à régler exigent des prises de conscience plus élaborées, plus concertées, mieux mises au point que l'affrontement systématique d'un côté ou de l'autre. Et enfin, c'est la garantie pour tous les grands courants politiques du pays, c'est-à-dire pour tous les citoyens, d'être représentés à mesure de leur engagement et de leur vote. Et je veux vous rappeler, je veux rappeler à votre groupe, qu'à la libération, lorsque le général de Gaulle était était à la tête des institutions du pays, le mode de scrutin qu'il a choisi, c'est la proportionnelle. Et peut-être pourrait-on réfléchir à tous ces facteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui monsieur le premier ministre et force est de constater que ça n'a pas été concluant puisqu'en 1958 le même général de Gaulle est revenu sur ce mode de scrutin. Rappelez qu'ici au Sénat, monsieur le Premier ministre, et je le dis avec la même amitié, c'est un mode de scrutin départemental et que les plus petits départements ont un mode de scrutin majoritaire. Et puis parce que je sais que vous aimez les grands auteurs, permettez-moi de conclure en citant Alain qui disait la représentation proportionnelle est un système évidemment raisonnable et juste, seulement partout où on l'a essayé, Elle a produit des effets imprévus et tout à fait funestes par la formation d'une poussière de partis dont chacun est sans force pour gouverner mais très puissant pour empêcher. C'est ainsi que la politique devint un jeu des politiques. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Stéphane Voisin pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. J'avais la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mes chers collègues. Avec ma collègue Viviane Mallet, également sénatrice de La Réunion, nous attirons votre attention sur l'aggravation de la situation sanitaire de Lille. Depuis plusieurs mois, La Réunion traverse une crise sanitaire préoccupante, marquée par une récrudescence rapide de l'épidémie de chinkungunya. Chaque jour, le nombre de cas graves augmente, alimentant l'inquiétude de la population et mettant en péril un système de santé déjà fragilisé. Samedi dernier, le décès d'une personne récemment vaccinée a conduit à suspendre la vaccination pour les plus de 65 ans. Cette décision a ravivé une méfiance déjà forte contre ce vaccin, compliquant encore davantage la mise en œuvre d'une réponse de santé publique efficace. Pourtant, des stratégies alternatives éprouvées ailleurs offrent des perspectives concrètes, fondées sur des approches biologiques innovantes. Ces méthodes mériteraient d'être sérieusement étudiées et surtout soutenues par le gouvernement. C'est notamment le cas du programme Volbakia qui pourrait servir aux Antilles et en Guyane. Ce programme, déployé avec succès en Nouvelle-Calédonie en 2019, a démontré son efficacité dans la lutte contre la dingue en agissant sur les moustiques aïdes égyptiques. Parallèlement, la technique de l'insecte stérile TIS qui cible les moustiques tigres aïdes albopictus représente une autre solution prometteuse pour des territoires comme la Réunion et Mayotte. Dans l'immédiat, des mesures simples mais fortes peuvent être engagées sans délai. La distribution gratuite de répulsifs anti-moustiques dans les zones à risque, la fabrication de moustiquaires en associant les communes et les CCAS, tout comme la suspension des jours de carence pour les personnes contaminées, relèverait à la fois du bon sens et d'un engagement en faveur de l'équité sanitaire. Mais au-delà de la réponse d'urgence, il est impératif de renforcer durablement nos infrastructures de santé. Aujourd'hui, elles sont au bord de la rupture. Monsieur le ministre de la Santé et de l'accès aux soins, ma question est donc la suivante. Quelles mesures concrètes, à court, moyen et long terme, le gouvernement tente-t-il prendre pour prévenir la progression de cette épidémie et soutenir nos concitoyens dans cette épreuve ? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, monsieur le ministre. Monsieur le dér. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Foissin, je crois que la lutte contre l'épidémie chikungunya est un combat partagé et collectif par tous, que ce soit naturellement les élus locaux de l'île, les élus nationaux ou naturellement le gouvernement. Cette lutte, vous l'avez dit vous-même, elle nous oblige, elle nous impose une mobilisation de chaque instant. par une mobilisation anti-vectorielle avec une mobilisation de près de 200 agents de l'agence régionale de santé, 250 militaires et de 800 PEC. Nous avons également l'utilisation dans le bouclier qualité prix de répulsifs pour pouvoir naturellement se protéger et puis de protéger les plus vulnérables et notamment je pense aux jeunes mamans et surtout aux nouveaux-nés puisque vous savez que dans les trois premiers mois de vie, les bébés sont particulièrement fragiles. Donc c'est la distribution de moustiquaires et puis naturellement la vaccination avec les risques que ça incombe et j'ai naturellement une pensée particulière pour l'ensemble des patients, des victimes du chikungunya et pour malheureusement le patient décédé dont l'imputabilité est possible vis-à-vis du vaccin qui nous a fait prendre des mesures de précaution conformément aux recommandations de la haute autorité de santé pour pouvoir protéger au mieux la population. Ce que je veux simplement vous dire, je suis allé moi-même visiter le Sirois pour justement voir si les moustiques stériles pouvaient être un élément de lutte important. C'est possible, on pourra envisager la commercialisation de ces moustiques à partir du mois de juillet. BPI est sur le sujet, l'Agence de l'innovation en santé également, pour éviter comme malheureusement, ou surtout pour ne pas éviter comme en 2005 ou 2006, où l'année supplémentaire, il avait été enregistré encore plus de décès. Donc je crois que c'est une mobilisation de tous de tous les instants pour soulager notre système de santé et prendre soin des compatriotes qui sont de la Réunion et qui sont fortement impactés par le chikungunya et par le cyclone récent. Non. La parole d'Etat, notre collègue Marie-Claude Lhermitte pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et chers collègues, ce qui se passe chez ArcelorMittal dans le Nord, à Dunkerque et sur les autres sites est une gifle. Des centaines d'emplois supprimés, des fonctions délocalisées, des salariés et leurs familles plongées dans l'angoisse de l'incertitude. C'est brutal et c'est inacceptable. Je leur exprime ici tout mon soutien, mais je suis sûre aussi du soutien des élus du territoire élargi, qui n'oublie pas que l'arrivée de ce fleuron de l'industrie, de ces salariés et de leurs familles, a permis le développement de nombreuses communes. Cette entreprise a été et est soutenue, accompagnée, défendue par l'État, la région et les élus locaux très investis. Aujourd'hui, elle licencie massivement avec peu de scrupules. Mais ce n'est pas seulement une trahison locale. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir de l'acier en Europe, un secteur stratégique que l'on veut soutenir et voir compétitif, décarboné, modernisé et renforcé.

Qui fixe réellement ces conditions et surtout quelles sont-elles ? Les salariés ont le droit de savoir, nous aussi. Ils sont toujours autant volontaires, prêts à se battre pour leur outil de travail qui fait leur fierté pour leur industrie verte, forte et compétitive. mais ils veulent des engagements clairs et réciproques. Alors, Monsieur le Ministre, quelle nouvelle garantie de l'usage efficace de l'argent public pouvons-nous exiger ? Quel cap clair pour l'acier, pour nos usines et pour nos emplois ? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de l'Industrie et de l'Energie, Monsieur Ferracchi. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Sénatrices, Madame la Sénatrice Marie-Claude Lhermitte. L'annonce par Arcelor de la restructuration qui va amener à la suppression de plus de 600 emplois sur 7 sites en France dont celui de Dunkerque est évidemment une mauvaise nouvelle et mes pensées vont aux salariés, à leurs familles, Je sais l'angoisse que fait naître ce type d'annonce et l'Etat, avec l'ensemble des services concernés, seront évidemment mobilisés pour accompagner socialement le reclassement de ses salariés. Mais au-delà, vous avez raison de mentionner, Madame la Sénatrice, que ce qui se joue, c'est l'avenir de la filière sidérurgique en France et en Europe. Cette filière, elle est soumise à des tensions très fortes. La production d'acier en Europe a baissé de 20% entre 2018 et 2023. On le sait, cette production est soumise à une concurrence féroce, une concurrence souvent déloyale, notamment de la part de la Chine, qui subventionne massivement ses producteurs d'acier, comme elle subventionne d'ailleurs massivement beaucoup d'autres filières industrielles. Par rapport à cela, les réponses ne peuvent pas être uniquement au niveau français, elles doivent être au niveau européen, c'est la raison pour laquelle Nous nous sommes engagés, le gouvernement et moi-même, à faire des propositions qui ont été reprises il y a déjà quelques semaines par la Commission européenne et en particulier des propositions qui visent à assurer une meilleure protection commerciale de notre industrie sidérurgique avec des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire des quotas à l'importation renforcés. Ces clauses rentreront en vigueur dans quelques temps. Vous me demandez qu'est-ce qui détermine les investissements dans la décarbonation et en particulier les investissements à Dunkerque. Il se trouve que j'ai rencontré hier la direction d'Arcelor. Elle est venue à Bercy et j'étais en ligne avec la direction Europe d'Arcelor. Il m'a été précisé très clairement que pour investir, et nous sommes tous d'accord sur le fait que pour maintenir l'emploi, il faut que ces investissements se fassent, il faut plus de protection commerciale. Il faut des coûts de l'énergie compétitif et nous y travaillons dans le cadre des négociations qui ont lieu avec EDF. Et il faut un soutien aux investissements. L'État y est prêt et tous les investissements qui seront soutenus ne le seront qu'à qu'à partir du moment où les dépenses sont effectivement engagées. Voilà nos engagements et vous dire encore une fois que nous sommes convaincus de l'absolue nécessité de soutenir cette industrie de souveraineté qui est l'acier sur notre territoire. Merci. Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous rappeler l'idée émise de mettre tous les protagonistes autour de la table. Vous savez pouvoir compter sur l'engagement et le soutien de tous les élus du territoire. Merci. La parole est à notre collègue Ahmed Lawedge pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président. le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, notre pays affronte une crise sanitaire silencieuse mais profonde, celle de la pénurie médicale. Dans un contexte de multiplication des déserts médicaux, nous avons aujourd'hui une solution concrète et immédiate. Des praticiens à diplôme hors Union européenne. Ces médecins, présents depuis des années dans nos hôpitaux et nos cabinets, sont pleinement engagés. Ils exercent avec compétence, souvent dans des conditions difficiles. Je reprends ici vos propres mots, Monsieur le Ministre, lorsque vous dites que beaucoup de nos services tiennent aujourd'hui grâce au pas dû. Ils sont reconnus par leur chef de service et leur chef de pôle. À l'occasion des épreuves de vérification des connaissances sur près de 4000 postes initialement annoncés, seulement 3044 postes ont finalement été ouverts. Ainsi, de nombreux candidats pourtant brillamment admis aux épreuves se retrouvent aujourd'hui écartés. 20% des postes ouverts restent vacants. Un constat alarmant qui souligne l'absurdité de la situation. Des médecins compétents et indispensables restent sur la touche alors que les déserts médicaux s'étendent chaque jour davantage. Monsieur le ministre, vous avez promis une simplification de leur parcours. Mais pourquoi attendre 2026 ? Pourquoi reporter une réforme alors que ces praticiens compétents sont disponibles immédiatement dans l'urgence sanitaire que nous connaissons ? Je vous demande donc très concrètement Pourquoi ne pas agir sans délai, par décret ou voire réglementaire, pour valider l'intégration de ces médecins, indispensable à nos territoires ? Je souhaite conclure mon intervention en y associant mon collègue Jean Yves Roux, très engagé sur ces sujets de santé dans les territoires. Et je veux remercier chaleureusement les médecins présents aujourd'hui dans les tribunes. Leur engagement mérite notre reconnaissance, mais surtout notre action. Merci pour vous répondre. La parole est au ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, monsieur Noderre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Lwadj, vous avez raison et je partage beaucoup de ce que vous avez dit. Effectivement, les déserts médicaux sont une des principales préoccupations de nos concitoyens. C'est pour ça que le Premier ministre a souhaité, dans le Cantal, faire un certain nombre de déclarations et laisser un certain délai assez court pour pouvoir proposer des solutions rapides dès le mois de septembre. Le seul point de désaccord, monsieur le sénateur, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Ça passera par une formation initiale augmentée, ça passera par le fait de récupérer nos étudiants français qui sont partis étudiés à l'étranger, comme en Roumanie, en Espagne ou Belgique, et ça permettra d'installer nos docteurs juniors dans de bonnes conditions. Concernant les PADU, effectivement, il ne faut pas avoir l'hypocrisie de ne pas reconnaître leur travail. Ils représentent 30 à 40% de certains de nos effectifs d'hôpitaux et ils assurent une grande partie de l'offre de soins sur notre territoire. dès 2025 puisque effectivement nous allons simplifier par voie réglementaire la voie interne qui va nous permettre effectivement de mesurer leur connaissance mais les compétences vont être assumées et mesurées localement par les médecins, chef de service, chef de pôle, président de CME et ça dans le souci de simplification ça sera fait dès 2025 et ensuite pour passer d'un mode de concours

qui nous permettra de porter cette simplification attendue par tout le monde, particulièrement par les Français pour se faire soigner. Je vous remercie. remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous parlez de simplification de concours, mais le problème est immédiat et concret. Permettez-moi de vous citer l'exemple de ce chirurgien urologue en poste à l'hôpital Cochin. Il a obtenu 18 deux moyennes en théorie aux épreuves des EVC. Il est d'ailleurs soutenu par le président de l'association française d'Urologie. Allons-nous sérieusement demander à un médecin de ce niveau, déjà en fonction de repasser son concours ? Ce n'est pas de simplification future dont nous avons besoin. C'est un décret immédiat pour valider qui ont réussi à occuper dès maintenant les postes vacants dans les déserts médicaux. La santé des Français ne peut plus attendre.

je prends aujourd'hui la parole devant vous au nom du groupe socialiste pour vous dire notre douleur face à l'assassinat d'Aboubacar Sissé. pour vous dire aussi que nous saluons le changement de position de la présidence du Sénat, qui, ce matin, disait qu'une minute de recueillement était une hystérisation du débat et qui s'y est rendu. Monsieur le Président, vous avez eu raison. Une minute de recueillement est toujours du baume sur les cœurs, du baume sur les âmes, et vous avez eu raison de changer de position. Il y a, monsieur le ministre, mes chers collègues, devant la barbarie, un vertige. Un vertige qui s'est propagé dans tout le pays puisque dans tout le pays, des rassemblements républicains, des rassemblements citoyens sont venus dire non aux crimes qui avaient été commis. Ils sont venus aussi dire non à ce qui était pressenti sous ce crime. Parce que s'il y a bien sûr toujours un mystère du mal de celui qui assassine, il y a un contexte dans lequel le mal se produit. Et ce contexte aujourd'hui, c'est celui du conditionnement progressif de la société française à la détestation des musulmans. Il est des éditorialistes tous les jours, tous les jours, pour affirmer que l'islam est incompatible avec la République. Il est des influenceurs tous les jours et la semaine dernière dans l'Oise sur les réseaux sociaux pour dire que le nom et le prénom des médecins qui nous soignent est trop arabo-musulman pour eux. Il est des essayistes pour discerter sur une idée empoisonnée le fait qu'il y aurait désormais deux peuples et non un peuple sur le territoire de la République. Et il est hélas, et je dis bien hélas, des ministres de l'Intérieur qui se sont laissés aller qui se sont laissés aller à des propos d'estrade, à des propos d'estrade, disant qu'il fallait mettre à bas la pratique cultuelle de centaines de milliers de femmes musulmanes dans notre pays sans faire la distinction, sans faire l'indistinction entre celles qui exercent leur liberté de conscience et celles et celles qui sont forcées de le faire. Ma question elle est simple, ma question elle est simple. Monsieur le ministre, est-ce que nous pouvons enfin compter sur vous ? Pour répondre, la parole est à nos ministres auprès du ministre d'État et ministre de l'Intérieur, François Noël Buffet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Je connais trop cette maison pour savoir que le propos doit être mesuré et qu'il ressort Et qu'il est Et qu'il est absolument nécessaire que, ici et singulièrement ici au Sénat, chacun mesure les enjeux qui sont devant nous et l'importance des mots qui sont utilisés. Le crime qui a été commis dans le Gard la semaine dernière et qui a tué Aboubacar Cissé est un crime barbare inacceptable. Je ne reviens pas sur les faits puisque chacun les connaît et que nous avons tous bien conscience de cette abominable situation. La seule information que je puisse vous donner cet après-midi, c'est que l'auteur s'est rendu à la police italienne, accompagné d'un parent et d'un conseil, et qu'il a accepté évidemment de revenir en France et que son retour en France est prévu pour la mi-mai. Il sera naturellement jugé et il est vrai que le procureur de la République compétent a indiqué qu'il percevait probablement un certain nombre de signes d'actes racistes mais naturellement l'enquête judiciaire qui est ouverte nous permettra d'en savoir plus. Quant au reste, la position du gouvernement comme celle du ministre de l'Intérieur, comme la mienne aujourd'hui et comme à l'une à l'imiter je l'espère bien de cette maison, est à la modération dans le propos, car nous sommes sur un chemin glissant. Un certain nombre d'élus, nationaux ou pas nationaux, de personnalités, de quelque nature que ce soit, jettent dans notre pays le poison de la division, et évidemment le poison d'un communautarisme insupportable. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. J'ai dit J'ai dit que j'en reprends pas dans la polémique, mais tout de même, un certain nombre de personnalités utilisent fortement ce moyen-là à des fins, finalement, électoralistes, je le dis, et de mauvais sens. Mais, mais, mais, mais... Faut conclure. Mais, j'indique. Mais oui, monsieur le Président, je conclue sur ce mot. Ce qui doit être le plus important, c'est l'unité nationale, l'unité absolue, rassemblée autour de nos valeurs, que quel que soit le banc que nous occupons, soit parfaitement défendu, et le gouvernement y veillera. veillera. La parole est à notre collègue Sylvana Silvani pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. À l'automne dernier, ArcelorMittal a annoncé la fermeture de ses sites de Reims et de Denain. En février, la direction française du groupe confirmait la délocalisation de 150 emplois supports vers l'Inde. Les syndicats lucides y ont vu le signal d'une restructuration plus lourde et ils avaient raison. Aujourd'hui, c'est une saignée industrielle qui est engagée. 636 emplois supprimés dans les coqueries et assieries du groupe à Dunkerque, Mardic, Dèvres, Bassindre, Mouson, Montaterre, Florange. Et pendant ce temps, ArcelorMittal engrange les profits. 36 milliards d'euros depuis 2019, près de 12 milliards de rachats d'actions pour satisfaire ces actionnaires et 298 millions d'euros d'aides publiques rien que pour l'année 2023. Une situation d'autant plus indécente que l'acier est au cœur de toutes les transitions. Dans le ferroviaire, les énergies renouvelables, la construction, les équipements industriels, partout où l'on veut produire, transformer, bâtir, le métal est là. Monsieur le Ministre, Sans compter les victimes collatérales, comme les travailleurs de la centrale d'ECASIS à Dunkerque. Il y a 15 000 salariés en France qui s'inquiètent pour leur avenir et de l'horizon de la taxation de l'acier carboné en 2030. D'où ma question. Afin de garantir la pérennité des emplois et des savoir-faire, que comptez-vous faire pour contraindre pour contraindre ArcelorMittal à engager la décarbonation des sites, quitte à faire évoluer la législation pour contraindre au remboursement des aides publiques perçue par le groupe. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de l'industrie d'énergie, monsieur Ferracchi. maintenir la production d'acier sur notre sol, sur le sol français est une absolue nécessité, je veux le dire et le rappeler. Dire également que Les salariés qui sont concernés par cette restructuration, qui sont au nombre de plus de 600, sont aujourd'hui dans l'angoisse, leur témoigner du soutien et dire que les services de l'Etat seront évidemment à leurs côtés pour accompagner la restructuration. Il est évident que nous devons agir pour pérenniser la construction et la fabrication d'acier sur notre territoire. Que devons-nous faire ? Nous devons d'abord travailler collectivement avec l'ensemble des acteurs. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les élus concernés par les restructurations. les restructurations sur l'ensemble des sept sites qui ont fait l'objet d'annonce de la part d'Arcelor. J'ai eu l'occasion d'échanger hier avec la direction d'Arcelor au niveau français et avec la direction d'Arcelor au niveau européen. Et pour répondre à votre question, Madame la Sénatrice, ce qui ressort de ces échanges, c'est que pour engager les investissements qui sont absolument nécessaires à la pérennité de nos emplois, nous devons agir sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est celui de la protection commerciale. C'est celui de la protection commerciale. Le deuxième levier, c'est celui des coûts de l'énergie. Et nous y sommes extrêmement sensibles. avec les négociations qui ont lieu aujourd'hui avec EDF. Le troisième levier pour engager les investissements en matière de décarbonation, ce sont les aides. Je veux vous le dire madame la sénatrice, il n'y a pas d'aide qui soit versée, que ce soit à Arcelor ou à d'autres entreprises, sans contrepartie. Les aides ne sont versées qu'en contrepartie de la réalisation d'investissements, qu'en contrepartie de la réalisation de dépenses, et sans ces investissements, les aides sont reprises. C'est la raison pour laquelle les 850 millions d'euros d'aide qui ont été mis sur la table par l'Etat, s'agissant des investissements d'Arcelora-Dunquerque, n'ont pas été versés parce que les investissements n'ont pas été réalisés. Je veux vous dire que nous avons l'intention d'agir sur tous ces leviers. L'ambition, c'est de pérenniser l'ensemble des sites afin d'éviter la fermeture de ces sites en France. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, l'Italie et le Royaume-Uni ont repris le contrôle de leurs aciéries et vous. Vous continuez de croire au mythe du marché autorégulateur. Il ne s'agit pas de nationaliser dans la débâcle pour revendre dans la prospérité, mais de faire de la propriété publique un outil de planification, de transition et de souveraineté. Prise de participation, fonds souverains livrés pour la réindustrialisation, baisse drastique des quotas européens d'importation de l'acier asiatique, les outils existent. Ce qui manque, c'est la volonté de rompre avec cette impuissance organisée. La parole est au président Guillaume Gontard pour le groupe Ecologie Solidarité. Pardonnez-moi. La parole est à madame Christine Herzog pour le groupe de l'Union centrale. Pardonnez-moi, c'était le même sujet. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, croyez-vous en la fatalité ArcelorMittal vient d'annoncer un plan national de suppression de 600 emplois en France, dont 200 en Florent-Jeune, en Moselle. La délocalisation des gens entamés des fonctions supports vers l'Inde et la Pologne et l'arrêt de l'investissement du groupe sidérurgique dans un outil productif laisse craindre un désintérêt de sa part pour la production d'acier en France. Et pour cause. Arcelor Mittal a retardé son projet d'acier décarboné dans l'usine de Dunkerque alors qu'il fait partie d'un contrat passé avec l'Etat. Et Arcelor Mittal n'investit plus dans le train à florent Jean Mauzel sous outil de production d'acier. Au contraire, celui-ci a investi massivement en Inde et au Brésil dans des usines modernes qui fonctionnent selon un cahier des charges environnementales moins contraignant que celui imposé par les normes européennes, car il veut rester compétitif dans l'économie mondiale. Nous sommes Nous sommes félicités, monsieur le ministre, de la transition énergétique de la centrale à charbon de Saint-Avold vers du biogaz, alors qu'au même moment l'aide, l'Inde pardon, serait juissée d'atteindre un record de production d'électricité à partir du charbon. Alors que l'acier en France est en crise, que le coût de la main d'oeuvre est élevé, que l'énergie coûte très cher et que les objectifs environnementaux à atteindre sont très contraignants pour les entreprises. L'Etat doit agir, entamer des négociations pour convaincre ArcelorMittal de rester en France et pour connaître ses projets. Monsieur le ministre, va-t-on sacrifier notre souveraineté si chirurgique à dire adieu à nos savoir-faire en laissant totalement et fatalement la France perdre son industrie si tel est le cas La nationalisation de l'entreprise est-elle une question sur la table ? Quelle est, monsieur le ministre, la version stratégique de l'État pour sauver notre souveraineté sidérurgique ?

Il n'y a pas de fatalité, y compris pour des filières en difficulté comme notre filière sidérurgique. Il n'y a pas de fatalité lorsque nous sauvons la Syrie à Châtilly-Driou, à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Il n'y a pas de fatalité lorsque nous sauvons les fonderies de Bretagne, il y a encore quelques jours à Caudan dans le Morbihan. Je crois profondément qu'en agissant sur les bons leviers, en se battant collectivement avec l'ensemble des élus, on peut obtenir des résultats et on peut garantir ce que vous appelez de vos vœux et ce que nous appelons de nos vœux, à savoir le maintien de notre souveraineté industrielle sur cette filière absolument essentielle, qui est nécessaire à tous les autres, car l'acidérurgie et l'acier est absolument indispensable à beaucoup de filières qui sont en aval, comme l'automobile, comme la défense. Les négociations, les discussions avec Arcelor, elles ont déjà commencé. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai échangé hier avec la direction d'Arcelor pour comprendre les raisons de cette décision et pour comprendre surtout les perspectives et la stratégie d'Arcelor en France et en Europe. Vous le savez, les difficultés de la filière sédérologique, elles ne sont pas que françaises. Thyssen Group en Allemagne a annoncé 11 000 suppressions d'emplois avec des fermetures de sites il y a encore quelques semaines. En France, aujourd'hui, aucun site ne ferme. Notre responsabilité, est que cela reste un objectif et qu'aucun site ne ferme à l'avenir en France. C'est l'objectif que nous poursuivons et pour cela nous devons agir, vous l'avez dit, dans plusieurs directions. D'abord en protégeant mieux nos industries. Nous avons des objectifs en termes de décarbonation. Ces objectifs, ils doivent être aussi les objectifs et les contraintes que nous faisons peser sur les exportateurs chinois qui envoient de l'acier en Europe. C'est l'objectif de la révision du mécanisme de taxation carbone aux frontières que nous portons et que la Commission européenne, par la voix du commissaire Céjournay, a reprise dans son plan d'urgence pour l'acier le 19 mars. Nous devons également agir, vous l'avez dit, sur les coûts de l'énergie. Nous espérons que d'ici au 1er janvier 2026, avec la fin du système de la Rennes, un certain nombre de contrats qui sont aujourd'hui en négociation entre les industriels électro-intensifs, dont Arcelor et EDF, vont se conclurent. Je suis pour ma part confiant sur le fait que nous arriverons également à lever cette contrainte. La stratégie, elle s'appuie sur plusieurs leviers, la compétitivité, la protection, et nous devons sortir d'une forme de naïveté à cet égard. Je vous remercie. La parole est cette fois-ci à Guillaume Gontard, Président pour le groupe écologiste Solidarité et territoire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. Vendredi 25 avril, à Boubacar-Sisset, fidèles musulmans étaient mortellement poignardés à 40 reprises dans une mosquée en croyant transmettre le rite de prière à son infâme assassin. Merci Monsieur le Président d'avoir changé d'avis et d'avoir concédé un moment de recueillement, c'était important. Car de la profanation d'un sanctuaire maculé du sang d'un innocent, à la duprie haineuse de l'assassin, tout, tout dans cet acte est profondément révoltant. À la famille et aux proches d'Aboubacar VI, nous adressons nos condoléances les plus émus. Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi des mots justes pour qualifier l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé vendredi. Vous avez également entendu aussi la souffrance, la peur et le sentiment de relégation exprimés par nos compatriotes musulmans depuis vendredi. Ce sentiment partagé sur nos bancs que les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le ministre de l'Intérieur et des cultes, n'ont pas exprimé une émotion à la hauteur du supplément de violence symbolique que représente l'assassinat d'un fidèle dans une mosquée. le sentiment que les plus hautes autorités de l'État n'ont pas pris la mesure de la gravité inouïe de cet attentat. L'histoire de France comme celle du monde nous enseigne qu'aucune guerre de religion n'a jamais rien produit d'autre que de la haine et de la désolation. La France en a tiré la conclusion la plus exemplaire qui soit en inventant la laïcité, définie dans la loi de tolérance et de liberté de 1905. Monsieur le Premier ministre, vous en avez justement rappelé hier à l'Assemblée nationale un principe fondamental, la loi protège la loi. Qu'allez-vous donc faire pour que cesse, notamment au sein du gouvernement et des émissiques parlementaires, cette instrumentalisation incessante de la laïcité pour stigmatiser l'islam et les musulmans ? Qu'allez-vous faire pour lutter réellement contre la montée de l'islamophobie avant que d'autres drames ne surviennent ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Gontard. je puis vous assurer que que la totalité des responsables publics actuellement au sein de l'exécutif, et je le crois, au sein de nos assemblées, partage la même certitude. Celle que vous avez exprimée, que j'ai moi-même défendue dans plusieurs livres sur les guerres de religion, que là est un démon jamais endormi. Il y a là un danger perpétuel qui ne cesse de se réveiller et singulièrement dans les temps de crise. Et ce danger, il s'articule très simplement, très clairement. L'autre est un ennemi. Or, nous croyons tous que vous avez rappelé la maxime que je cite souvent. La loi protège la foi mais la foi ne fait pas la loi. L'idée que non seulement la tolérance, j'ai écrit sur l'édit de Nantes comme vous savez, non seulement la tolérance mais au-delà de la tolérance, la compréhension mutuelle, l'idée que nous ne sommes pas des étrangers les uns aux autres, que nous avons à construire, j'ai dit hier, tous nos compatriotes musulmans, tous nos compatriotes juifs, tous nos compatriotes chrétiens, tous nos compatriotes agnostiques et nos compatriotes athées et d'autres tous ont droit de citer. Et j'ai ajouté hier qu'à mon sens, nous devrions creuser l'idée de devoir de citer. Nous avons le devoir de construire ensemble quelque chose qui est de la citoyenneté et du destin partagé. Le drame du Gard est épouvantable tellement, vous l'avez dit, il est entaché de tous les symptômes de ce que nous cherchons à combattre et de ce que nous devons décrire. Et je suis heureux de sentir l'unanimité qu'il y a en réalité sur ces bancs, sur cette détermination à mener ce combat et à construire une cité différente. Merci, monsieur le Président. La parole est à notre collègue Laurent Saumont pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, monsieur le Ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, la seule réelle prison est la peur et la seule vraie liberté de se libérer de la peur, disait Aung San Suu Kyi. Les agents de la pénitentiaire vont-ils devenir les prisonniers de la peur que veulent instaurer les terroristes sous couvert de l'étendard fallacieux de la défense des droits des prisonniers ? Parmi les agressions contre les agents de la pénitentiaire, on compte 66 agressions graves en 2023 à l'intérieur des établissements contre lesquels le ministère de la Justice agit. Mais depuis le 13 avril, comme à Saint-Quentin-Fallavier ou Villefontaine en Isère et dans 31 départements, on recense à ce jour plus de 60 faits criminels sur des établissements et plus grave encore sur des véhicules ou domiciles d'agents pénitentiaires comme à deux reprises à Amiens envers la même surveillance. Des faits d'intimidation, de nuisance, de destruction, de tir sur les domiciles, d'incendie, de tag avec la signature, défense des droits des prisonniers ou encore des messages cryptés envers les personnels ou leurs familles. Ce terrorisme est un défi lancé à notre République et à l'État de droit qui ne peut être toléré sous couvert de revendications grotesques de défense des droits de l'homme. Nous devons tous le condamner. Comment prétendre défendre les droits de l'homme et s'attaquer aux biens et menacer les personnels des administrations pénitentiaires eux-mêmes ? La lutte au sein des établissements contre la circulation de produits illicites, d'armes ou des moyens de commandité des exactions hors les murs démontre que les mesures prises sur les fouilles et les mesures adoptées avec la PPL narcotrafique au Parlement dérangent une organisation mafieuse, lucrative et meurtrière. Monsieur le Ministre, quelles consignes sont données au préfet pour garantir la sécurité des biens et des familles des agents pénitentiaires ? Et quelles mesures engagez-vous pour débusquer ces terroristes, redonner confiance et sérénité à nos fonctionnaires dans l'exercice de leurs missions ? Pour vous répondre, la parole est auprès du ministre de l'État et du ministre de l'Intérieur. Monsieur François-Noël Buffet, vous avez la parole. Évidemment que le problème que vous soulevez est un problème majeur et nous sommes déterminés à ce qu'il ne perdure pas. Mais vous avez raison de rappeler que depuis le 4 avril, plus de 150 actions ont été commises ont été commises à l'encontre des centres bénéficiaires ou de leur personnel sur l'ensemble de notre territoire. Je voudrais les citer. J'ai le cocktail Molotov sur le parking de l'École nationale de formation des agents à agents incendie volontaires devant la maison d'arrêt de Ville-Pinte. Rafal de Kalachnikov sur la prison de Toulon. des véhicules d'agents pénitentiaires brûlés, des surveillants pénitentiaires menacés, notamment à Amiens. Ces faits, qui sont des menaces, des intimidations, ces tirs de mortiers, constituent toute évidence une riposte au texte qui a été voté récemment, désormais définitivement et le tenons à vous en remercier puisqu'il participe et nous permet et permet au gouvernement de pouvoir continuer sa lutte contre le narcotrafique et ses effets néfastes. Rappelez que le gouvernement a pris immédiatement des dispositions de soutien et de protection des agents pénitentiaires dans le cadre d'un plan et de mobilisation à la fois du garde des Sceaux et à la fois bien sûr du ministre d'État de l'Intérieur. Dans la nuit du 15 avril, nous avons rejoint l'ensemble des préfets ainsi que les services de police et de gendarmerie placés sous leur autorité de renforcer de renforcer sans délai les mesures de protection à l'égard des personnes et des biens relevant de l'administration pénitentiaire. Le 15 avril, les préfets de zone, les services de police et de gendarmerie dont les services de renseignement et l'administration pénitentiaire ont été réunis pour conforter et préciser ces instructions. Enfin le 17 avril, une instruction commune définissant les modalités de renfort de renforcement de la sécurisation des sites et des personnels d'administration pénitentiaire exigeant une mobilisation forte et coordonnée a été diffusée.

pour vous indiquer que le Parquet national antiterroriste coordonne désormais l'ensemble des investigations. Des moyens importants ont été déployés pour identifier, rechercher et interpeller les auteurs, bien évidemment. À ce jour, plus de 30 interpellations ont déjà eu lieu dans toute la France et les gardes à vue, évidemment, des gardes à vue, pardon, sont toujours en cours. Je terminerai simplement pour dire que le gouvernement et ses moyens sont entièrement mobilisés pour protéger nos prisons, ses personnels, évidemment, leurs familles, car il ne peut pas en être d'ailleurs autrement. Merci. Laurent Saumon. Oui, messieurs les ministres, la peur doit changer de camp. La liberté, disait Montesquieu, est le droit de ce que les lois permettent, permettre aux personnels pénitentiaires de la peur, la libération conditionnelle à l'exercice serein et sécurisé de leur métier dont l'application de l'anonymisation de leur identité dans les procédures est une mesure cardinale. Merci. La parole est à notre collègue Audrey Inquilel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur Monsieur le ministre de l'Industrie, demain, 1er mai, la mobilisation sociale sera particulièrement forte dans les sites touchés par les 600 suppressions de postes annoncées par Ars et l'Hormital il y a quelques jours, dont 300 confirmées ce matin même pour le Nord. Pour Dunkerque et Mardic, comme pour Dèvres, Montaterre, Florence, Indre ou Mouson, nous serons nombreux demain à défiler, à témoigner notre solidarité aux salariés et aux élus qui s'inquiètent. Pourquoi ces suppressions de postes sur l'outil de production qui viennent s'ajouter aux plans sociaux déjà en cours sur les fonctions supports ? Pourquoi la suspension de ces investissements censés pérenniser l'activité et sur lesquels l'État s'est déjà financièrement engagé ? Pourquoi ce manque de transparence de la part d'un industriel aux résultats pas si mauvais et toujours demandeurs d'aide publique. Oui, le marché européen de l'acier souffrait depuis longtemps, mais la filière acier est essentielle et, à ce titre, elle est d'ailleurs soutenue au plan national et européen. Nos hauts fourneaux français et européens ne doivent donc pas être sacrifiés, ils doivent plus que jamais être électrifiés pour faire face aux enjeux énergétiques, économiques, écologiques et pour préserver notre souveraineté comme nos emplois. Si la décarbonation et la modernisation ne sont pas rapidement et directement assurés par ArcelorMittal, il faut que la France et l'Union européenne prennent de nouvelles mesures fortes pour garantir la production locale d'acier bas carbone par d'autres moyens, y compris l'entrée au capital ou la nationalisation temporaire des aciéries. Monsieur le ministre, en ce joli mois de mai, qui célèbre le travail, mais aussi une Europe née justement d'une communauté autour de l'acier, pouvez-vous auprès des salariés et de nos territoires prendre ici l'engagement concret que la France aura l'audace de tout faire avec ses partenaires pour que l'acier soit notre histoire et aussi notre avenir Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Lincolnel. Oui, la France est mobilisée. La France a été à l'initiative en Europe pour soutenir un plan d'urgence pour la sidérurgie européenne. J'ai convoqué à Paris un sommet le 17 février avec l'ensemble des ministres concernés par la production sidérurgique, avec l'ensemble des représentants des filières, avec les organisations syndicales, avec la Commission européenne, pour mettre sur la table un certain nombre de propositions visant à nous défendre. Je dis nous défendre parce que le sujet est bien celui de la défense. La défense face à une concurrence qui est déloyale, la concurrence en particulier de l'essai chinois, massivement subventionnée, très fortement carbonée dans sa production. Et vous l'avez dit, un des enjeux c'est la décarbonation. Donc nous agissons et nous agissons au niveau européen. Mais nous n'agissons pas qu'au niveau européen. Vous serez mobilisés demain, et je sais votre engagement, l'engagement de l'ensemble des élus, le maire de Dunkerque, Patrice Vergret, le président de la région, Xavier Bertrand, l'ensemble des parlementaires, et j'ai eu l'occasion de répondre à un certain nombre de questions sur le sujet, hier et aujourd'hui à l'Assemblée. Le travail ne peut être que collectif. Nous devons résoudre le problème de la protection commerciale et être très ambitieux. Nous ferons pression sur la Commission européenne et je rencontrerai, après avoir rencontré la direction d'Arcelor hier, le commissaire Stéphane Sejourné dans les prochains jours pour porter à sa connaissance l'ensemble des leviers que nous proposons pour que les investissements dans la décarbonation, que vous appelez de vos voeux, que nous appelons de nos voeux, se fassent. Pour que ces investissements se fassent, il faut agir sur la protection commerciale, il faut agir sur la taxation carbone aux frontières qui rentrera en vigueur aux promesses en 2020-2026 avec le souci que cette taxation soit efficace nous faisons des propositions pour qu'elles le soient. Il faut agir sur les coûts de l'électricité. Il faut agir sur tous les enjeux de compétitivité. Et vous le savez, l'État est en soutien de l'investissement de la filière cédiérurgique et de tous les industriels pour leur décarbonation. pour cela, il faut évidemment que les industriels prennent des décisions. Nous allons créer les conditions pour qu'ils le fassent. Nous le ferons avec l'ensemble des élus. Et je vous remercie également pour votre engagement sur ce sujet. Merci. La parole est de notre collègue Agnès Evreine pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur. Le 1er avril dernier, un maître de conférence a dû interrompre son cours à l'Université de Lyon 2 sous les huées et les injures de militants cagoulés et masqués. Cette intrusion, revendiquée par un groupuscule autoproclamé anti-France, est une triple agression. agression contre la liberté académique, contre la démocratie et contre la laïcité, évidemment. Vous-même, Monsieur le Ministre, avec la Ministre d'État, aviez annoncé votre soutien total au Professeur Balanche. Or, Monsieur le Ministre, qu'avez-vous nous vu depuis ? Une présidente d'université qui prend ses distances avec l'enseignant et dénonce des propos complotistes et délétères. Des collègues universitaires qui chipotent, malgré l'évidence ici, sur le fantasme d'un islamo-gauchisme. Et comme toujours, les Sampiternelles appellent au calme, dignes du traitement si triste et si célèbre du pas de vague. Alors, certes, l'indépendance de l'université est précieuse. Pour autant, les autorités universitaires ne sont pas au-dessus des lois et les universités ne sont pas des zones de non-droit, monsieur le ministre. Alors nous attendons une position sans ambiguïté du gouvernement. Ma question est très simple. Quelles sanctions ont été enclenchées contre ces militants qui ont ouvertement défié les lois de la République ? Je vous remercie. On vous répond. La parole est au ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Philippe Baptiste, vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci Monsieur Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Evren, je vous remercie pour votre question. Je veux tout d'abord effectivement confirmer le fait que le 1er avril, un maître de conférence de l'Université de Lyon 2 a été interrompu pendant son cours. C'est parfaitement scandaleux, c'est une situation honteuse qui ne devrait pas arriver. par des individus qui étaient des individus qui étaient masqués et nous lui avons apporté un soutien Je voudrais vous signaler aussi que la présidente de l'université a pris toutes les décisions à ce moment-là qui s'imposaient du soutien fonctionnel au dépôt de plaintes, etc. Elle a eu une expression malheureuse qu'elle a publiquement clarifiée après et elle a été après, à son tour, victime d'un acharnement qui lui aussi, madame, est injustifiable. Avec le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Rotailleau, nous avons dû nous assurer qu'elle bénéficiait comme Fabrice Balanche, le maître de conférence qui a été attaqué initialement de toutes les protections nécessaires. Il est intolérable que le maître de conférence, comme la présidente d'université, ait été menacé de mort pour simplement ces actions, enfin c'est scandaleux ce qui s'est passé dans cette université, et j'appelle effectivement, ce n'est pas pas de vague, c'est un appel à l'art retenu. L'université est un lieu de dialogue, est un lieu de confrontation intellectuelle, est un lieu de liberté académique qui doit être encadré par la loi, toute la loi et strictement la loi, Cela veut dire en particulier que nous serons extrêmement vigilants sur tous les débordements qui peuvent être de nature antisémite. Nous sommes aussi et nous travaillons aussi efficacement sur les sanctions qui peuvent être prises. par les étudiants ou par des personnels qui pourraient avoir à un moment ou à un autre débordé. Nous travaillons aussi étroitement avec le garde des Sceaux pour que tous les articles 40 qui concernent ces faits soient systématiquement traités. traités. Je voudrais simplement signifier que le cadre disciplinaire lui aussi est en train d'être simplifié et amélioré grâce à une PPL qui a été votée ici même au Sénat à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Écoutez, je n'ai pas entendu la réponse à ma question, notamment qui était très précise sur les sanctions. Je le rappelle, ce qui s'est passé à Lyon n'est pas un petit incident provoqué par des petits jeunes exaltés. C'est une affaire très grave. Je le rappelle et je le pense profondément. C'est une offensive concertée d'une extrême gauche intolérante et d'un islamisme qui teste tous les jours nos limites. il faut en finir avec cet équilibrisme et je le dis droit dans les yeux, il faut en finir avec cet équilibrisme et réagir avec célérité, avec clarté et avec force parce que nous n'avons que trop commenté la tête baissée et ça suffit. Maintenant il faut agir contre ce nouvel obscurantisme qui met à mal les fondements de notre université au-delà notre cohésion nationale. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Annick Billon pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Demain 1er mai, de nombreux artisans boulangers et fleuristes garderont le rideau baissé. Non par choix, mais par crainte d'être verbalisés. L'an dernier, 5 artisans vendéens ont été poursuivis. pour avoir pétri leurs pattes un jour férié. Le 25 avril 2025, le tribunal de police de La Roche-Churion les a finalement relaxés. C'est un soulagement, certes, mais le flou persiste pour l'ensemble de la profession. Face à cette incertitude juridique, le groupe union centriste s'est mobilisé sans attendre. Nous avons alerté la ministre du Travail dès le mois de mars, puis le 18 avril pour y associer les fleuristes également concernés. Pendant 20 ans, ces professionnels ont travaillé le 1er mai sans difficulté. Aujourd'hui, la situation est tubuesque. Un particulier pourrait vendre du muguet sur le trottoir, mais le fleuriste devrait garder boutique close. C'est pourquoi, avec le président Hervé Marseille, nous avons déposé une proposition de loi visant à préciser les établissements pouvant bénéficier d'une dérogation leur permettant d'ouvrir le 1er mai. Ce texte ne remet pas en cause ce jour férié et chômé. Il ne cherche pas à ouvrir une brèche mais à combler un vide juridique. Il ne banalise pas, il clarifie. La procédure accélérée a été engagée par votre gouvernement. Je remercie madame la ministre Catherine Vautrin pour son soutien. Toutefois, les professionnels sont dans l'attente. Deux questions, monsieur le ministre. La jurisprudence du tribunal de la Roche-Churion sécurise-t-elle les ouvertures de demain ? Et quel calendrier avez-vous imaginé pour faire aboutir notre texte ? Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Billon, Madame et Monsieur les Sénateurs, pardon, vous posez effectivement la question sur le travail du du 1er mai. Permettez-moi effectivement de vous le rappeler, mais vous le savez parfaitement, c'est la tradition française, le 1er mai est un jour férié, chômé et rémunéré. Et on peut difficilement dérogée à cette règle qui est celle du code du travail hormis les conditions que nous connaissons tous de maintien et de nécessité de services publics au public comme l'hôpital, les EHPAD ou tout un tas d'organisations qui sont jugées essentielles. Cependant vous posez la question d'une évolution du travail dans notre société Et votre étonnement est relativement compréhensif. Nous avons tous été sollicités dans nos surconscriptions par fleuristes boulangers qui souhaitent travailler. La législation en vigueur permet à chaque artisan boulanger de pouvoir travailler mais ne permet pas à ses salariés de le faire. Donc effectivement il faut peut-être envisager, je crois que nous sommes une société qui favorise le travail et de pouvoir permettre cette évolution législative sur la base du volontariat, de permettre aux boulangers, aux fleuristes d'ouvrir avec les salariés qui souhaitent les accompagner dans cette action. Donc c'est le sens de votre proposition de loi que vous avez faite, soutenue par le sénateur Hervé Marseille. Cet agenda sera naturellement à l'étude prochainement, ne réglera certainement pas le problème de demain d'ici quelques heures. Par contre, la ministre Panossian-Bouvet et la ministre Vautrin ont invité les artisans boulangers à se rapprocher de leurs organisations professionnelles, pour elles-mêmes se rapprocher vis-à-vis vis-à-vis des services de l'État pour éviter la situation que vous avez vous-même décrite. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Je remercie le gouvernement pour son soutien. Je remercie les artisans qui animent nos centres-villes et nos centres-bourges. Et j'espère que de nombreux Français et Françaises pourront acheter leur pain et leur mullet demain 1er mai. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Pascal Alizard pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les relations avec l'Algérie restent passionnelles, mais depuis plusieurs mois, se sont aussi bien dégradées. Ne faut pas se le cacher, si le régime algérien se redit à l'égard de la France, c'est parce qu'il nous sent impuissants et divisés. Comme nombre de Français, j'avais cru comprendre de l'engagement du président de la République et du gouvernement que les choses étaient plus apaisées, que la coopération reprenait et qu'allait s'enclencher une nouvelle phase de la relation bilatérale. La réalité est en fait bien différente. Placement en détention d'un agent consulaire algérien pour enlèvement et séquestration, expulsion réciproque, rappel de notre ambassadeur. Monsieur le ministre, face au blocage, face à la désinformation orchestrée ou encouragée, le gouvernement fera-t-il enfin preuve de davantage de fermeté ? Les accords franco-algériens dans le domaine de l'immigration sont un des leviers, il en existe d'autres. Cette frébrilité prendra-t-elle fin ? Et dénoncerez-vous l'accord de 1968 ? Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Alizar, je vous remercie de votre question. Vous le savez, sur ce sujet comme sur tant d'autres, notre seul boussole c'est de défendre les intérêts de la France et des Français. Nous avons souhaité avoir un dialogue exigeant avec l'Algérie, un partenariat d'égal à égal, pour défendre nos intérêts, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'Algérie respecte ses engagements au regard du droit international, pour reprendre ses ressortissants expulsés, pour reprendre la coopération dans les domaines de la défense, la sécurité ou encore du renseignement, et bien sûr pour obtenir la libération de notre compatriote, l'écrivain Boalem Sansal, injustement condamnés et emprisonnés aujourd'hui en Algérie. C'était le sens de l'échange téléphonique entre le président de la République et le président Teboun. C'était aussi, bien sûr, le sens de la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barreau, à Alger. Mais pour un dialogue, il faut être deux. Notre justice, justice indépendante, a pris la décision, vous l'avez rappelé monsieur le sénateur, d'arrêter des ressortissants algériens pour leurs activités en France. Face à cela, l'Algérie a eu une réponse totalement disproportionnée, injustifiée et brutale d'expulser 12 de nos ressortissants, 12 agents auxquels je voudrais d'ailleurs La La réponse de la France a été extrêmement ferme, en réciprocité. Nous avons expulsé 12 diplomates algériens et rappelé en effet notre ambassadeur. Sur ce sujet, notre position est très claire. L'Algérie décide de reprendre le dialogue et que nous pouvons ensemble défendre nos intérêts. Nous y sommes ouverts. Mais si l'Algérie fait le choix d'une relation dégradée, de l'escalade et de la crise, nous saurons y répondre. Et nous avons une palette de leviers et d'instruments, en effet, pour assumer un rapport de force et pour pouvoir nous défendre. Monsieur Alizar. Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse, un peu à complète puisque sur l'accord de 68 vous n'avez pas répondu. J'en prends acte. Rappelez quand même que le rapprochement par exemple, parce que c'est un des points de désaccord entre Paris et Rabat sur la question du Sahara Occidental, est un faux prétexte parce qu'il est plus d'ailleurs une conséquence qu'une cause de la dégradation des relations avec Alger et que ce rapprochement d'ailleurs s'inscrit dans un large mouvement international. Je note aussi que l'Algérie est un partenaire important de la Russie en Méditerranée, elle pourrait le devenir davantage aussi en raison de la perte d'influence russe au Levant, En Afrique francophone, la Russie aussi montre son savoir-faire et à chaque fois l'Algérie n'est pas très loin. Alors Monsieur le Ministre, compte tenu de l'attitude de plus en plus exigeante et intransigeante d'Alger, des actions sur notre territoire, du contexte international que je viens de rappeler, trop souvent basé sur le rapport de force, le temps est vraiment venu de faire passer des messages politiques sans ambiguïté. Isabelle Vriquet pour le groupe socialiste, écologiste et républicaine. Chers collègues, il y a huit ans, la majorité promettait mon merveille avec la suppression de la taxe d'habitation. Plus de pouvoir d'achat pour les Français, pas de paire pour les collectivités et des finances publiques sous contrôle. Mais aujourd'hui, les faits sont étus. Le déficit public atteint 5,8% du PIB, la dette publique dépasse 113% du PIB, Les collectivités locales sont privées de leviers fiscaux et dépendent des dotations de l'Etat. Le financement des services publics locaux est déséquilibré. Le Conseil est sans appel. Les collectivités locales, injustement accusées de dégrader les comptes publics, ne sauraient être des variables d'ajustement budgétaire, ni être quantonnées à un simple rôle de guichet de l'Etat. Pourtant, le président de la République continue d'exclure toute remise en question d'une décision déjà injustifiée en 2017, devenue en 2025 totalement irresponsable. Le ministre Reb Samen a récemment évoqué l'idée d'une contribution des citoyens au financement des services publics locaux. Cette proposition a le mérite d'ouvrir le débat sur la fiscalité locale et plus largement sur les ressources des collectivités. Vous êtes donc assez lucide pour mesurer l'impasse dans laquelle nous sommes. Alors, allez-vous continuer de défendre la suppression de la taxe d'habitation, réforme que vous savez au fond mauvaise, ou choisirez-vous de redonner aux élus locaux l'autonomie financière dont ils ont besoin ? Pour répondre, la parole est au ministre d'Aménagement du territoire de la décentralisation, François Rebsaben. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Madame la Sénatrice Isabelle Bricquet. Votre question va me permettre de mettre au point trois niveaux de réponse. Premièrement, la taxe d'habitation a été supprimée. Elle a été annoncée pendant la campagne électorale du président de la République, il a tenu ses engagements, il a supprimé la taxe d'habitation. Beaucoup de parlementaires aujourd'hui envisagent de rétablir, mais je n'ai vu aucune proposition de loi déposée par un parlementaire sur ce sujet. C'est la première chose. La deuxième chose concerne l'état de nos finances publiques. Nous sommes aujourd'hui, sous l'autorité du Premier ministre, en train de faire la pédagogie de l'état de nos finances publiques, c'est-à-dire du grave déficit qui frappe notre pays. Et je voudrais dire à cet égard que rien n'est arbitré mais que la pédagogie continue. Je recevrai mardi prochain l'ensemble des associations d'élus. Elles sont au nombre de sept, connues et reconnues. Et nous débattrons ensemble de réflexions sur les propositions qui pourront être faites dans le cadre de cette réflexion. Et rien n'est arbitré s'agissant du budget. Enfin, troisièmement, j'évoque depuis longtemps et je vais continuer à le faire. Je l'ai fait devant la délégation aux collectivités territoriales que préside le sénateur Bernard Delcroc. Je pense que nous ne pourrons pas durer longtemps avec un nombre de personnes qui financent les communes, à savoir les propriétaires. Dans certaines communes, il y a 30% de propriétaires et 70% de personnes qui ne payent pas l'impôt local. mon idée, mais ce n'est pas la seule, elle est reprise par la collectivité bien souvent, mon idée c'est qu'à terme, il y ait une contribution pour que chacun mesure les efforts de services publics qui sont faits par nos communes et qu'on recrée ainsi un lien citoyen entre le consommateur habitant et la municipalité et la municipalité qui exerce le pouvoir du service public. Vous c'est aussi une faute politique, faute pour les collectivités privées d'une grande part d'autonomie fiscale et financière, faute pour l'État qui perd chaque année plus de 20 milliards en compensation, et je crois que l'État n'en a pas besoin, et pour les contribuables locaux, vous venez de le préciser, Mais faudrait-il encore qu'une contribution s'évalue avec un niveau de revenu, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, et ça nourrit, vous le savez, l'eurosentiment. Faut conclure. Refuser conclure. Refuser de reconnaître cet échec, c'est condamner un peu plus nos collectivités, donc il faut agir. La parole est à notre collègue Pauline Martin pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Preuve de la ferveur des parlementaires pour défendre nos artisans. Alors en cette veille de 1er mai, à l'instar de ma collègue Annick Billon, il est difficile de faire l'impasse sur la polémique qui gronde en territoire. Demain, nos boulangers, nos fleuristes ne pourront pas laisser travailler leurs salariés en une journée par définition fleurissante pour ces secteurs. Mieux encore, le ministère va lui ordonner à ses agents de travailler afin de surveiller l'absence de travail. On marche sur la tête. Encore plus détonant, chacun pourra installer un étal afin de vendre quelques brins de muguets alors que nos commerçants devront faire grise mine. à l'heure où l'Etat invite les Français à travailler plus pour soutenir notre économie en berne et assurer nos retraites. Voilà que l'Etat lui-même empêche nos travailleurs d'exercer leur activité, privant ainsi les salariés, bien souvent volontaires, d'une rémunération bonifiée en ce jour férié, chômé et payé. Si le Code du Travail doit être respecté, je m'interroge sur la façon dont nous avons vécu cette vête du travail depuis 1948. Monsieur le ministre, sans attendre l'adoption d'un texte consensuel proposé par nos collègues, pourrions-nous envisager que vos inspecteurs profitent de cette journée ensoleillée pour acheter fleurs et baguettes sans contrôle ni verbalisation ? Monsieur le Président, madame et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Billon, je ne sais Pardon ? Même question, alors pas même réponse. Madame la sénatrice Martin, mes excuses. Vous avez mis beaucoup d'enthousiasme dans votre question. Je vais essayer d'y mettre autant d'enthousiasme dans la réponse pour vous dire que nous sommes totalement d'accord avec ce que vous venez d'évoquer. Le 1er mai est un jour férié, chômé et rémunéré. Cependant, le Code du travail, nous ne l'avons pas écrit aujourd'hui et si nous souhaitons tous collectivement le modifier pour permettre justement ces initiatives locales que vous saluez, J'ai les mêmes boulangers dans ma circonscription, les mêmes fleuristes que vous, eh bien il faudra modifier le code du travail. J'ai vu que, pardon, la sénatrice Billon en avait proposé, avait fait une proposition de loi. J'imagine vous-même également, et je crois que c'est... le Sénat qui va pouvoir examiner l'évolution, de pouvoir encourager le travail et je crois que nous partageons cette valeur du travail pour finalement saluer l'engagement de ceux qui se lèvent tôt le matin et qui veulent pouvoir contribuer à la croissance Cependant, vous savez qu'il existe déjà des situations d'exception. J'ai parlé tout à l'heure des hôpitaux, des EHPAD, on pourrait rajouter naturellement les sapeurs-pompiers. Vous avez entendu que je n'ai pas cité les agents du ministère de la Santé et du Travail qu'Astrid Pagno-Sanbouvet a demandé aux fédérations de boulanger de se rapprocher des services de préfecture pour éviter ces situations UBS que vous avez très bien décrits. Mais moi je crois en la sagesse du Sénat pour permettre une voie d'ouverture, pour permettre de travailler plus sur la base du volontariat et d'avoir une société française qui puisse s'adapter et qui puisse aussi se simplifier comme le souhaite le Premier ministre. Je vous remercie. Madame Martin. Monsieur le Ministre, vous l'avez compris, avant de compter sur nous, nous comptons sur vous. Bien. La parole est à notre collègue Eric Dumoulin pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre Montchalin, chers collègues. On vient de l'évoquer, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation vient de lancer ce qu'on pourrait appeler un ballon d'essai sur la création d'une sorte de nouvel impôt local, une contribution modeste demandée à tous les ménages pour le financement des services publics des communes. Au-delà du buzz médiatique, cette annonce s'apparente en réalité au rattrapage d'un péché originel, celui de la suppression de la taxe d'habitation. mal réfléchis, mal financé, cette réforme a profondément déstabilisé tous les défis déjà fragiles des finances locales. Par ce jeu de bonnes taux fiscales, les communes et par ricochet les départements ont perdu toute ou partie de leur autonomie. Profondément déstabilisée et pourtant incomparablement plus vertueuse que l'Etat, elle souffre. Accessoirement, on l'a vu, cette réforme aura coûté environ 20 milliards au budget de l'État, ce qui ne l'aide pas aujourd'hui à combler son abyssal déficit. La fiscalité locale repose donc désormais sur les seuls propriétaires. Les locataires ne financent plus les services publics de proximité, dont ils sont pourtant bénéficiaires au quotidien. Cette distorsion contribue à créer un fossé entre les citoyens d'une même ville. Faut-il également rappeler que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public et que dans un contexte de crise et de très faible croissance, elles constituent pour le tissu économique et les entreprises une ressource absolument vitale. Il convient donc de les protéger, de les accompagner, plus que de les ponctionner à l'aveugle. S'il est compréhensible qu'elles participent à l'effort national de redressement des comptes publics, elles ne peuvent devenir la variable d'ajustement trop facile des comptes ou plutôt des mécontes de l'État. Elles sont à ce jour profondément inquiètes de ce que l'État leur concocte pour le budget 2026. les chiffres d'un doublement voire d'un triplement de l'effort demandé en 2025 hantent les couloirs. Donc Madame la Ministre, dans l'attente d'une grande réforme et d'une indispensable remise à plat de tout le système de financement des collectivités locales, je n'aurai qu'une seule question. Que pouvez-vous leur dire pour les rassurer et nous rassurer ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la Ministre chargée des comptes publics, publics, Madame de Montchalin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, pour vous rassurer et pour vous répondre, d'abord je veux être très clair, ce gouvernement ne souhaite pas instaurer dans le prochain budget de nouveaux impôts et nous sommes le pays record du monde des impôts et nous avons, je crois, une très grande fierté dans ce gouvernement d'avoir pu rendre 700 euros en moyenne aux Français par la suppression de la taxe d'habitation. Le deuxième élément de ma réponse, c'est qu'à moyen terme, et le ministre Ebsamen l'a dit, Le lien entre le contribuable et le service public, le lien entre le citoyen et son maire, sont des choses sur lesquelles nous pouvons probablement donner plus de visibilité et de clarté à l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, je fais le lien aussi au niveau national pour que les Français comprennent mieux, voient mieux où vont leurs impôts. Troisième élément, comment nous allons travailler pour ce projet de loi de finances de 2026 pour les collectivités ? Mardi prochain, le premier ministre Eric Lambert et moi-même allons lancer la conférence de financement des territoires qui a un objectif, redonner de la prévisibilité aux collectivités. Le grand malentendu aujourd'hui, c'est que d'abord, effectivement, les collectivités ne sont pas les filales de l'État. Mais le grand malentendu, c'est qu'un maire, il est élu pour six ans, et moi, ministre des Comptes publics, je fais le budget sur un an. Et cette dichotomie, cette désynchronisation de nos agendas crée beaucoup de malentendus. Les maires veulent savoir où ils vont et l'État doit lui être garant de notre retour à 3% de déficit en 2029. Comment y arriver ? Par le dialogue, la co-construction, la remise en question des normes trop nombreuses qui créent des dépenses inutiles, par la réflexion sur nos ressources humaines, sur la fonction publique territoriale, sur le pilotage par les maires eux-mêmes et par les collectivités de leurs dépenses, et donc nous allons co-construire une trajectoire pluriannuelle et un cadre de prévisibilité. Je pense que c'est une manière mature dans le dialogue, dans les faits, de regarder comment collectivement, en étant solidaires des finances de la nation, nous revenons ensemble à une situation où nous ne créons pas de dettes supplémentaires pour nos enfants. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous en avons terminé. Merci Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres. Je vous rappelle, nos prochaines questions d'actualité auront lieu le 7 mai. La séance sera reprise à 16h30 pour le débat sur le rapport d'avancement annuel sur le plan budgétaire et structurel. Madame la Ministre, de moyen terme, 2025-2029, très bon 1er mai, n'oubliez pas, les baguettes et le muguet. La séance est suspendue.

L'asséance est reprise. Prenez place, chers collègues. Bonjour Madame la Ministre. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010 prise pour son application, la Commission des affaires économiques a mis un avis favorable, 20 voix pour, 4 voix contre, à l'anomination de M. François Jacques aux fonctions de président du Conseil d'administration du Centre national d'études spatiales. Un avis défavorable, 14 voix pour, 28 voix contre, à la nomination de M. Bernard Fontana, aux fonctions de président directeur général d'Electricité de France. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à aménager le Code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale ont été publiés.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 C'est une demande de la Commission des Finances. La parole est tout de suite à madame la ministre chargée des comptes publics. Madame de Montchalin, vous avez la parole. Je vous en prie Madame la Ministre.

cher Sénateur, Mesdames et Messieurs les Sénatrices, il y a désormais trois mois, le Parlement a adopté le projet de loi de finance pour 2025, issu, nous le savons, d'un compromis trouvé en commission mixte paritaire. Ce compromis nous oblige à un suivi renforcé de l'exécution de ce budget afin de respecter les équilibres financiers qui ont été trouvés par vous, parlementaires, au premier rang duquel notre objectif de déficit de 5,4 %. Alors ce suivi d'exécution est d'autant plus nécessaire que les aléas et les risques sont décuplés, nous le voyons cette année, sous l'effet de la double crise que nous traversons, la crise géopolitique et la crise commerciale. Dans le cadre du rapport annuel d'avancement, nous venons ainsi, aujourd'hui, vous rendre compte du respect de notre trajectoire de rédressement des comptes publics, à commencer par le respect de notre cible de déficit pour 2025, et c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter les principes de construction du budget 2026. Ce rapport annuel d'avancement que nous présentons aujourd'hui comporte deux volets. D'abord les constats et ensuite les corrections. C'est-à-dire les aléas et les risques d'une part et d'autre part les mesures de correction pour tenir notre trajectoire. C'est le sens de la méthode du « quoi qu'il arrive » que nous avions pu vous présenter non seulement lors de la Commission des finances qui s'était réunie et nous avait auditionné il y a quelques semaines, mais également il y a deux semaines lors du premier comité d'alerte. La loi de finances initiale pour 2025 a déjà engagé un effort courageux dans le sens du redressement de nos finances publiques en s'appuyant sur un budget de compromis. L'objectif de 5,4% de déficit est, et je cite ici la Cour des comptes et le Haut Conseil aux finances publiques, un objectif impératif, ambitieux et atteignable. Pour nous y tenir, vous le savez, nous avons déjà mis en place une gestion renforcée qui a pu donner lieu à trois circulaires du Premier ministre, qui concerne notamment les reports de crédit qui ont d'ores et déjà été strictement réduits. Je rappelle que les reports généraux hors relance du budget général ont été réduits de moitié pour 4,4 milliards entre 2024 et 2025 désormais. D'autres mesures conservent, vous le savez, la réserve de précaution qui était désormais sanctuarisée au niveau interministériel de 8,7 milliards. Par ailleurs, nous avons aussi lancé, et c'est une nouveauté, une gestion prudentielle de Londam. Catherine Vautrin, vous le savez, a constitué, avec toutes les équipes qui sont en charge des dépenses de santé, une réserve effective de 1,1 milliard d'euros. Et par ailleurs, vous l'avez vu, deux circulaires du Premier ministre concernant l'une l'efficience hospitalière et l'autre le suivi resserré de la masse salariale de l'État. Mais face aux nouveaux aléas géopolitiques, économiques et financiers dont Éric Lombard vous parlera, nous avons été amenés, ainsi que d'autres économistes, à réviser notre prévision de croissance pour 2025 à la baisse à 0,7% plutôt que 0,9%. En conséquence, comme je vous l'avais annoncé lors de votre audition en commission des finances, face à des risques avérés, nous avons pris des décisions, notamment celle de nous redonner des marges de prudence à hauteur de 5 milliards d'euros sur l'État, ce qui représente 0,6% des crédits ouverts en loi de finances. C'est donc un effort à la fois substantiel mais tout à fait atteignable. Ces 5 milliards portent pour moitié sur une annulation de crédit qui avait été mise en réserve dont le décret a été publié en fin de semaine dernière et comme nous l'avons transmis au président et au rapporteur général, ce sont 3,1 milliards en autorisation d'engagement et 2,7 milliards en crédit de paiement qui ont été annulés et ne seront donc pas consommés. Ces crédits, vous le savez, proviennent pour l'essentiel de la réserve de précaution initiale dont le taux avait été fixé comme en 2024 à 5,5% et pour lesquels il avait été demandé instamment au ministère de ne pas compter sur ces crédits dans leur programmation je peux parler ainsi, anticipée. L'autre moitié de l'effort pour les 5 milliards porte sur un surgel ciblé des crédits afin de reconstituer nos marges qui a été lui aussi abouti en ce début de semaine. Ce sont 2,8 milliards de crédits qui ont ainsi été mis de côté de nouveau pour reconstituer notre mise en réserve initiale et qui pourront, le cas échéant, si la conjoncture venait à se dégrader ou si de nouveaux risques venaient à émerger, de que nous puissions de nouveau les annuler. Nous ferons, comme nous nous sommes engagés, un deuxième point d'étape sur le suivi de l'exécution fin juin lors d'un deuxième comité d'alerte. Et comme lors de ce premier comité, nous vous ferons connaître en toute transparence l'intégralité des informations dont nous disposons, que ce soit sur les recettes que nous collectons, sur les dépenses, leurs trajectoires et toutes les mesures nécessaires à prendre pour tenir les équilibres financiers de la loi de finances initiale. En deuxième sujet à aborder avec vous, je voudrais vous présenter quelques orientations pour le budget 2026, d'ailleurs appelé autour du Premier ministre le 15 avril dernier. Pour nous, un des premiers prérequis pour que nous arrivions à reconstruire ensemble un compromis comme nous l'avons fait cet hiver, c'est bien, je le redis, de tenir et de maîtriser nos dépenses publiques dès cette année et ensuite de fixer un certain nombre de principes que je crois chacun de nos concitoyens, et vous ici au premier chef, pourront partager. Le premier principe, c'est de redire que nous devons absolument faire en sorte que les dépenses, en particulier de fonctionnement, ne progressent pas plus vite que la croissance économique. Cela peut sembler une tautologie. Néanmoins, aujourd'hui, dans de nombreux domaines, nous observons que depuis plusieurs années, voire parfois plusieurs décennies, il y a eu des hausses de dépenses supérieures à la croissance et ainsi une génération automatique de déficit. Cela doit concerner aussi bien l'État que la sécurité sociale ou les collectivités territoriales. Par ailleurs, deuxième principe, nous le savons, un certain nombre de subventions publiques sont aujourd'hui perçues comme des droits acquis par un certain nombre d'acteurs, des ménages, des entreprises, des associations ou des collectivités. Et à ce titre, les subventions de l'État ont donc perdu ce que j'appellerais leur effet déclencheur. Elles sont parfois devenues des effets d'aubaine. Par conséquent, c'est bien l'efficacité de la dépense publique qui a été réduite. L'État, à nos yeux, doit planifier et agir efficacement plutôt que de se contraindre à n'être qu'un guichet. C'est bien l'exercice qu'a annoncé le Premier ministre de refondation de l'action publique qui doit nous conduire à réinterroger l'action de l'État et de ses opérateurs pour que, chaque fois, nous agissions quand c'est nécessaire et non pas quand cela est une habitude. Troisième principe, c'est celui d'une exigence là aussi tout à fait démocratique. Nous ne pouvons redresser économiquement le pays si nous n'arrivons pas à ce que les intérêts particuliers se mettent en retrait face aux intérêts généraux, face à l'intérêt général de la nation. Il faut ainsi que nos choix budgétaires puissent refléter plus clairement des objectifs politiques clairs et que nous acceptions de réformer aujourd'hui ce qui nous aidera demain. Cela peut aboutir, et nous devons je crois ici le partager et l'assumer, à ce que des pertes pour certains à court terme puissent être acceptées si elles se font au bénéfice de la croissance et du gain-don pour des millions d'autres citoyens à terme. Quatrième principe, il est essentiel que nous puissions mettre fin à certaines dépenses qui ne sont plus aujourd'hui justifiées. Je pense en particulier à des coûts liés à la redondance et à l'enchevêtrement des compétences et des responsabilités. Je pense aussi à des dépenses qui ont trop fortement augmenté depuis la crise sanitaire, telles que les arrêts maladies. Et enfin, il est essentiel que nous puissions faire toute transparence sur le coût et la valeur des services publics qui sont trop souvent méconnus de nos concitoyens pour qu'ils redonnent un sens à leurs impôts et aux bénéfices qu'ils retirent de la dépense publique. Ces objectifs, ces principes, devraient nous permettre de construire ensemble un budget qui fasse du sens et qui nous permette de tenir notre trajectoire, de revenir sous les 3% de déficit en 2029 en commençant par une première marche à 4,6% en 2026. En parallèle, nous avons une méthode, la transparence totale, pour que les parlementaires puissent avoir toutes les informations nécessaires pour suivre l'exécution de ce compromis et surtout pouvoir jouer pleinement leur rôle constitutionnel nous évaluer et plus largement évaluer nos dépenses publiques, nos finances publiques. Et à ce titre, vous le savez, nous pensons que le printemps de l'évaluation sera un moment important et utile pour nous tous pour que cette trajectoire de reprise en main soit une trajectoire partagée. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à monsieur Eric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

monsieur le rapporteur général du budget, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, j'ai l'honneur de vous présenter au nom du gouvernement et aux côtés de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, l'état d'avancement de notre plan stratégique. budgétaire à moyen terme, le PSMT, qui permet d'établir une perspective sur plusieurs années afin de proposer une trajectoire progressive, équilibrée, soutenue et suivie. Sur le point économique, comme vous le savez, nos prévisions de croissance ont été revues dans le cadre d'un contexte géopolitique que je qualifierais de tourmenté, ce qui est une litote. Le sénat de croissance est relativement proche que celui du projet de loi de finances du mois de janvier sur le plan domestique. Car, comme le montrent les dernières enquêtes de conjoncture, elle a relativement bonne tenue de la consommation des ménages. L'adoption du budget en 2025 a permis de réduire l'incertitude. Cependant, la dégradation de l'environnement international amène à revoir à la baisse, notre prévision de croissance pour 2025, à 0,7%, c'est-à-dire 0,2 points de moins que lors de notre scénario révisé du mois de janvier. C'est à la fois une conséquence de la politique tarifaire américaine et plus généralement de l'aléa qu'elle provoque. On a vu dans un chiffre qui vient de sortir que la croissance américaine a été légèrement négative au premier trimestre, ce qui est une mauvaise surprise En revanche, une assez bonne surprise pour notre pays. La croissance a été de 0,1% au premier trimestre, ce qui est conforme à ce qui était attendu. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que l'acquis de croissance sur 2025 est de 0,4%. ce qui fait que ce sera un combat et nous le conduirons, mais cela renforce notre objectif de 0,7 %. L'incertitude économique évidemment a fait que nos entreprises dégradent non seulement leur exportation, mais également leur niveau d'investissement. Au total, l'environnement l'environnement international pèserait sur la croissance à hauteur de 0,3 points contre 0,1 point également négatif anticipé en janvier. Cette incertitude engendre une aversion au risque accrue avec des mouvements significatifs ces derniers temps sur les bons du trésor et notamment sur l'écart de taux avec notre voisin allemand, même si les choses se sont un peu améliorées ces derniers jours. Pour ce qui est de nos finances publiques, Notre trajectoire de dépenses primaires nette a été amendée par rapport à celle proposée par la France dans notre PSMT d'octobre 2024. Il s'agissait de prendre en compte le changement de cible de déficit du gouvernement pour 2025 qui, comme vous le savez, est passé de 5% à 5,4% et de la recommandation émise le nouveau cadre budgétaire européen induit à un nouvel indicateur que je viens d'évoquer, le niveau de croissance de la dépense primaire nette, c'est-à-dire hors coût coût du portage de notre dette. Ce nouvel outil est plus précis que l'indicateur traditionnel de déficit public qui est particulièrement sensible aux élèves de conjoncture. Ainsi, le taux de croissance cumulé de nos dépenses primaires nettes reste identique sur la période 24-29 à celui qui était proposé dans le PSMT initial. D'ailleurs, on commule sur la période 24-25, la dépense primaire naître primaire naître croîtrait de 4,2 %, soit un niveau inférieur au maximum fixé par le Conseil à 4,6 %. Ainsi, la trajectoire prévue dans le nouveau cadre de gouvernance européen est bien suivie. Cela me permet de réitérer notre engagement à faire passer notre déficit sous la barre des 3 % en 2029. ce que le Premier ministre appelait très justement, lors de sa conférence de finances publiques, le seuil d'indépendance, le seuil d'indépendance de la nation naturellement. Pour satisfaire cet engagement, 3 % en 2029, nous maintenons notre objectif de 4,6 % de déficit en 2026, comme nous nous y étions engagés à l'automne dernier. Nous faisons ce qu'il faut, et la ministre vient de le rappeler, pour éviter le risque de dépassement de dépenses. Elle vous a présenté les 5 milliards d'euros d'économies. Nous nous sommes nous sommes déjà donné rendez-vous au mois de juin pour un second comité d'alerte et pour faire un point d'étape devant vous de l'exécution de votre budget 2025. Dans sa conférence de presse sur les finances publiques du 15 avril, le Premier ministre a confirmé une nouvelle méthode, celle d'un dialogue poussé entre le gouvernement et la représentation nationale, la Commission des finances, les représentants des élus et les partenaires sociaux. Cela doit nous permettre de partager les exigences qui est la nôtre de redressement des comptes publics et d'identifier ensemble les voies et moyens dont poursuivre la bonne réalisation. En effet, le retour à un niveau de déficit public soutenable n'est pas seulement une priorité budgétaire, c'est une priorité politique pour notre gouvernement. C'est aussi une priorité pour notre crédibilité à l'international, la garantie de notre souveraineté, et aussi cela permettra de continuer à libérer l'investissement, encourager les entreprises et l'emploi. Je vous remercie de votre attention et nous allons, avec la ministre, écouter attentivement réactions et commentaires. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à monsieur Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des Finances. Vous avez dix minutes, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, présenté il y a maintenant deux semaines en Conseil des ministres, ce premier rapport d'avancement annuel doit être transmis aujourd'hui même à la Commission européenne. plan budgetaire et structurel de moyen terme, le PSMT 2025-2029. Comme celui-ci, il est une nouveauté prévue par le nouveau cadre de gouvernance économique de l'Union européenne, entré en vigueur il y a un an, le 29 avril 2004. Je rappelle que ce PSMT, adopté en Conseil de Ministres le 23 octobre 2024 et dont le Sénat a débattu en séance publique le 30 octobre dernier, a été validé par le Conseil de l'Union Européenne le 21 janvier 2025. Sa trajectoire de dépenses avait toutefois été rectifié en janvier de cette année pour prendre en compte l'évolution de la cible du déficit 2025 entre les gouvernements Barnier et Bérou et à cet instant je veux quand même préciser que le Sénat n'a pas eu connaissance à l'époque du détail de cette révision. J'en viens à mon analyse du rapport d'avancement à proprement parler en débutant d'abord par un point sur la situation économique de notre pays. Entre la fin 2019 et la fin 2024, le PIB de la France a progressé d'1,5 de moins que celui de la zone euro. tenter de se rassurer en constatant qu'il a augmenté de 4 points de plus que celui de l'Allemagne, mais dans les comparaisons, personnellement, je qualifierais de médiocre les performances économiques de la France depuis 6 ans. S'agissant des prévisions de croissance, le gouvernement revient dans ce rapport d'avancement assez fortement, d'ailleurs sur le scénario du PSMT 2025-2029, qui a été présenté fin octobre, alors que celle-ci s'est levée au départ à 1,1 %, elle est désormais de 0,7 %, ce qui met la prévision du gouvernement en ligne avec les autres prévisions officielles. Vous voyez qu'en moins de six mois, Il y a eu deux révisions. Une révision à la baisse qui résulte, certes, de la hausse des incertitudes que le gouvernement impute pour l'essentiel dans l'environnement international. Et malgré le recul des 04 points de croissance, il n'est pas exclu, il faut se le dire, que celle-ci puisse continuer à diminuer en raison notamment d'un certain nombre d'aléas négatifs. Cette orientation à la baisse se manifeste par le fait que les prévisions les plus récentes sont aussi plus pessimistes parfois que celles du gouvernement. Ainsi, la prévision de croissance du FMI pour la France, en date de la fin du mois d'avril, est aujourd'hui à plus 0,6%, de même que la prévision du consensus des économistes. La prévision d'avril de l'OFCE s'élève quant à elle à 0,5%. En gros et en résumé, je pense que les facteurs de croissance identifiés par le gouvernement pourraient être légèrement moins porteurs que s'ils envisagent Et peut-être que les facteurs de recul seront un peu plus marqués, mais je mets tout ça au conditionnel. D'après le rapport d'avancement, la croissance serait principalement portée par la consommation des ménages à hauteur de plus 1,2%. hors administration, alors qu'une progression même très limitée était envisagée en janvier par le gouvernement, l'investissement poursuivrait sa baisse malgré l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE et engagée depuis le printemps 2024. Pour le gouvernement, l'investissement des ménages reculerait de 0,3 points, celui des entreprises de 0,8. Ainsi, la demande intérieure privée hors stock contribuerait, selon le gouvernement, à hauteur de 0,5 points de croissance du PIB en 2025, en retrait minime de 0,1 points par rapport à la prévision gouvernementale de janvier. Si l'on suit les prévisions par contre du consensus économiste ou de l'OFCE, cette demande pourrait contribuer légèrement moins à la croissance, là encore ce qui paraît assez cohérent avec les prévisions du FMI. Cet écart qui d'ailleurs peut s'expliquer par une prise en compte limitée par le gouvernement, des effets de l'incertitude qui continuent à régner au niveau national. si on regarde l'OFCE, par exemple, pour l'OFCE, l'incertitude nationale grèverait la croissance de 0,3 points en 2025 et de 0,1 en 2024 et, conjuguée à une incertitude internationale grandissante, la situation politique toujours instable et le manque de visibilité sur les mesures de politique économique et fiscale renforcerait ou risque d'enforcer les comportements attentifs des entreprises. Les conditions de dégradation du marché de l'emploi, du ralentissement de l'activité, ça se manifeste évidemment, et on le sait, par une augmentation du chômage, aujourd'hui qui approche les 8% selon la Banque de France et le FCE, ce qui peut là encore freiner les comportements de consommation. Si on regarde la consommation publique, Quand elle, elle soutiendrait davantage la croissance qu'initialement prévue du fait d'une consolidation budgétaire moins marquée entre le début de la discussion du budget 25 par le gouvernement de Michel Barnier et la cible qui a été finalement retenue. Enfin, selon le gouvernement, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait nulle, à la différence de janvier. En janvier, c'était plus 0,1. Elle pourrait même être, si on suit l'OFCE, de moins 0,1. Tout ça est assez, comment dirais-je, réduit en tous les cas dans les perspectives. Ce recul est néanmoins une composante de l'assombrissement global du tableau de l'économie mondiale, résultant notamment et principalement de la politique commerciale américaine dont les effets seront, qu'on le veuille ou non, globalement négatifs sur l'économie française, l'augmentation des droits de douane que les États-Unis ont engagé en février 2025, renforcé le 2 avril, mais finalement compte tenu le 9 avril pour de nombreux pays dont la France pourrait grever selon le gouvernement la croissance de 0,3 points en 2025. D'ailleurs cette estimation ne prend en compte que les mesures annoncées jusqu'au début avril, jusqu'au 2 avril. Elle est par conséquent donc peut-être un tout petit peu surévaluée. Au total, les prévisions de croissance qui sont retenues dans le rapport d'avancement pour les années à venir sont donc révisées légèrement à la baisse, ce qui constitue de mon point de vue un scénario un peu plus réaliste qu'un maintien pur et simple des prévisions initiales du PSMT. Cette moindre croissance rendra assurément plus difficile l'atteinte du déficit et de la cible de déficit pour 2025. Revenons au dérapage majeur en 2023 avec, je le rappelle, un déficit de 5,4 points de PIB. La dégradation s'est poursuivie avec un niveau de 5,8 points en 2024 au lieu des 4,4% prévus dans la loi de finances pour 2024 et est dans la loi de programmation des finances publiques arrêtée fin 2023. La cible était alors de 3,7% pour le déficit public en 2025. C'est inscrit dans la loi de programmation des finances publiques. Elle est aujourd'hui, disons-le, complètement hors d'atteinte. Pourtant, la LPFP n'a que 18 mois d'existence. Je ne répéterai donc jamais assez que ces deux années de dégradation, 2023 et 2024, sont finalement terribles pour l'économie française. Elles sont inacceptables, mais elles sont inacceptables car elles sont injustifiables par la seule situation économique du pays ou par une quelconque crise, crise, comme je l'ai dit par rapport aux comparaisons européennes. Je pense qu'il est grand temps que les responsables politiques de l'époque cessent de continuer à clamer l'excellence de leur pilotage des finances. Je vous le dis, Monsieur le Ministre, les Français ne comprennent pas cette dérobade qui confine, et je le dis sans ménagement, à l'irresponsabilité. Je rappelle que pour l'année en cours, le gouvernement prévoit un déficit de 5,4 points du PIB. C'est quand même, par rapport aux prévisions de la loi de programmation des finances publiques, un écart de 50 milliards. L'ambition d'un retour du déficit à son niveau de 2023 reste atteignable. L'annulation de 2,7 milliards d'euros en crédit de paiement par le décret du 25 avril et la mise en réserve complémentaire d'un montant comparable qui est évoqué nous permettent de penser que le déficit et l'objectif est atteignable. Je vais terminer simplement en vous disant que globalement, l'engagement au niveau européen autour de la trajectoire de dépenses primaire net, qui est également notre trajectoire de correction dans le cadre de la procédure pour déficit excessif, est pour l'instant tenue. En 2025, l'évolution de cette DPN, prévue à plus 0,9, serait donc de 0,1 point supérieur à ce que recommande le Conseil, ce qui constitue un écart inférieur au 0,3, toléré par les nouvelles règles. Cette bonne orientation ne doit néanmoins pas nous faire perdre de vue, à la fois la nécessaire vigilance et le volontarisme qui doivent demeurer les maîtres mots de l'action publique en matière de finances publiques et pour nos comptes publics pour les années à venir. Je vous remercie. et merci. Monsieur le Président, madame et monsieur les ministres, monsieur le rapporteur général de la Commission de finances, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues, à la différence du dernier programme de stabilité que nous avons examiné en avril 2024, le rapport d'avancement annuel de cette année est, si l'on peut dire, de meilleur augure, même s'il hérite une situation de finances publiques très dégradée. Souvenez-vous, l'an dernier, alors que la loi de programmation avait été adoptée 4 mois plus tôt seulement, le programme de stabilité actait déjà sa caducité. Le dérapage de la cible de déficit par rapport à la loi de programmation est d'ailleurs massif en 2025 à hauteur d'environ 50 milliards d'euros. Cette année, le document dont nous débattons donne à voir effectivement un spectacle différent. La trajectoire de dépenses nettes qui nous engage au niveau européen, est tenue. La prévision de déficit pour 2025 est certes moins ambitieuse que dans le programme de stabilité mais n'éloigne pas trop, on s'en éloigne pas trop et demeure là même que dans l'article liminaire de la loi de finances pour 2025. Cela s'explique probablement davantage par la contrainte apportée par les nouvelles règles budgétaires européennes que par la seule vertu propre de ce gouvernement. Mais si elle existe sans doute, puisque s'écarter trop franchement de la trajectoire de dépenses nettes, qui est également pour nous la trajectoire de correction dans le cadre de la procédure de déficit excessif, se traduirait par des sanctions. Pour autant, je ne me réjouis pas trop vite. Si le rapport d'avancement annuel pour 2025 est un exercice de suivi du PSMT, il est aussi, d'une certaine manière, un exercice d'actualisation de prévision pour l'année en cours, puisque nous ne sommes qu'à la fin de son premier tiers. Or, la prévision de croissance pour 2025, actuellement de 0,7%, ne cesse de reculer. depuis six mois et on est en droit de se demander, même si vous êtes restés optimistes, monsieur le ministre, si ça ne reculera pas davantage, encore au gré des décisions et volte-face du président américain notamment. Le SMI prévoit une croissance de 0,6% pour la France. L'OFCE envisage 0,5%. Il est donc à craindre, on ne le souhaite pas, qu'on fasse un peu moins bien que prévu, que les recettes soient en retrait par rapport à la prévision et que le déficit soit en revanche légèrement plus élevé. Dans ces conditions, la revalorisation de la prévision de rendement de certains impôts me paraît imprudente. En particulier, la prévision d'impôts sur les sociétés pour 2025 a été revue à la hausse de 2 milliards d'euros en raison de résultats meilleurs qu'attendus en 2024. ce qui, selon moi, représente un risque qu'il ne semble pas opportun de prendre alors même que la prévision de rendement de cet impôt est toujours particulièrement incertaine du fait notamment du cinquième à compte. C'est devenu pour moi un leitmotiv que d'alerter sur ces incertitudes qui entourent toujours la prévision de l'impôt sur les sociétés qui appellent plutôt de manière générale à la prudence. En résumé, je constate que les chiffres du rapport sont bien dans les clous de ce que prévoyait le PSMT, mais qu'il est encore bien trop tôt pour affirmer avec certitude qu'on en sera au même point pendant toute l'année. Je précise ici que si la trajectoire de dépenses net effective se révélait conforme à celle qui était initialement prévue, cela s'expliquera pour l'essentiel par les mesures nouvelles en recette adoptées dans le budget 2025. Ce qui, au passage, valide la position que je défends depuis longtemps. Un redressement des comptes publics ne peut en aucun cas passer uniquement par une diminution de la dépense publique, du moins quand on est dans ces sommes-là. mais doit impérativement s'accompagner d'un volet recette. Je rappelle ici que le cumul des mesures en recette prises depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République représente une perte annuelle de plus de 60 milliards d'euros. Or, les mesures nouvelles en recette du budget 2025 étaient pensées pour être temporaires. Et c'est là que ce rapport d'avancement qui indique une volonté de faire des économies de 110 milliards d'euros d'ici à 2029 et reprend le projet du gouvernement d'en faire 40 milliards dès 2026, m'interpelle un peu et me rend sceptique voire méfiant. Il faut dire qu'on a des raisons depuis quelques années. Bien que ce nouveau document n'ait pas la même vocation prospective, à moyen terme que les anciens programmes de stabilité, je m'interroge sincèrement sur la capacité de ce gouvernement à tenir pour l'année prochaine et les années à venir ces engagements sans toucher aux recettes. Comment est-il possible de mettre fin à des mesures temporaires en recette tout en faisant des économies de 110 milliards d'euros en moins de 50 Peut-être pourrez-vous, Madame, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur ce point. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame Elisabeth Douano, rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales. Vous avez cinq minutes Madame la rapporteure générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Depuis la réforme du pacte de stabilité de l'année dernière, ce plan d'avancement annuel se substitue au programme de stabilité. Dans le cas des finances sociales, le rapport d'avancement se traduit par un recul important de l'information disponible pour le Parlement par rapport à celle figurant dans les programmes de stabilité. J'ai déjà d'ailleurs souligné ce point dans le cas du PSMT lors de notre débat du 30 octobre dernier. J'espérais que le rapport d'avancement permettrait de corriger cette lacune. Ce n'est malheureusement pas le cas. En effet, les programmes de stabilité comprenaient dans les annexes un tableau indiquant pour chaque année jusqu'à la fin de la programmation la capacité de financement prévisionnel par sous-secteur, c'est-à-dire en particulier pour les administrations de sécurité sociale. Ces données n'étaient pas disponibles sur le périmètre plus restreint de la sécurité sociale, mais c'était déjà ça. Cette programmation à moyen terme du solde des administrations de sécurité sociale n'existe plus ni dans le PSMT, ni dans le rapport d'avancement annuel. Certes, comme le souligne le Haut Conseil des finances publiques, le rapport d'avancement annuel se différencie des anciens programmes de stabilité en se voulant, dans l'esprit du législateur européen, un rapport de suivi du PSMT. En conséquence, il peut ne porter que sur les années passées et en cours. Il s'agit à mon avis toutefois d'un recul majeur de l'information du Parlement dans le domaine des finances sociales. D'autant plus dommageable qu'il n'existe aucune programmation des finances sociales. La loi de programmation des finances publiques de décembre 2023 a été caduque à peine voté et les tableaux pluriannuels annexés aux lois de financement de la Sécurité sociale ne sont que des prévisions à droit constant qui prévoit donc une aggravation du déficit de la Sécurité sociale. Je souhaite donc, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, vous poser la question suivante. Voyez-vous de réintroduire dans les prochains rapports d'avancement la répartition du besoin de financement prévisionnel entre sous-secteurs d'administration publique qui figurent dans les programmes de stabilité ? À défaut, serait-il possible de réintroduire une telle répartition dans un autre document, comme le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances ? Le rapport d'avancement comprend toutefois quelques informations relatives aux finances sociales pour les prochains exercices, en particulier dans son tableau de la page 56, soyons précis. Dans le cas de la réforme des allègements généraux, le tableau mentionne la prochaine mise en place d'un comité de suivi placé auprès du Premier ministre. Ce comité de suivi a en effet été instauré par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat. Ce comité doit publier un rapport avant le dépôt de chaque PLFSS, du PLFSS pour 2026 au PLFSS pour 2030. Pouvez-vous, Madame, Monsieur le Ministre, nous indiquer où en est la mise en place de ce comité de suivi ? Toujours dans le cas de la réforme des allègements généraux, le tableau de la page 56 indique que le gouvernement ne souhaite pas en rester à la réforme de la loi de financement de sécurité sociale pour 2025 et juge nécessaire d'aller plus loin. Il indique en effet, et là je vous cite, le gouvernement reste déterminé à réaliser une réforme globale des allègements généraux. Tout en garantissant la soutenabilité des comptes des administrations et de la sécurité sociale, cette réforme renforcera l'efficacité du dispositif des allègements généraux de cotisation sociale et encouragera également la mobilité salariale et la productivité pour les travailleurs rémunérés autour du SMIC. Pouvez-vous nous indiquer ce que le gouvernement a concrètement l'intention de faire ? Merci Merci madame la rapporteure générale dans la suite du débat la parole est maintenant monsieur grégory blanc pour le groupe écologie solidarité et territoire vous avez cinq minutes cher collègue Monsieur le président monsieur le ministre madame la ministre chers collègues S'il est un point qui caractérise les différents gouvernements depuis la sortie des crises Covid, c'est la constance. Pour ne pas dire l'entêtement, à afficher un discours musclé d'un côté et à agir à l'inverse dans les faits. Ainsi, il est tout à fait paradoxal de voir la succession des propos sous les gouvernements d'Elisabeth Borne à celui de François Bayrou qui s'inscrivent tous dans la même doxa fiscale de non augmentation des impôts, c'est le discours, et dans les faits le taux de prélèvement obligatoire continue d'augmenter. Ce décalage, ce paradoxe, pose un problème d'efficience dans la gestion, parce qu'en bloquant idéologiquement tout débat global, même pragmatique, et donc des réformes structurelles sur les recettes, vous empêchez dans les faits l'État d'être plus efficace dans l'impact économique et plus juste en termes d'égalité devant l'impôt. Votre approche qui consiste à faire à bas bruit le contraire de vos discours confine en quelque sorte à la schizophrénie. Finalement, ceux qui ont largement bénéficié de l'aide de l'État pendant le Covid n'auront pas à renvoyer l'ascenseur. Ce phénomène est créateur de tensions dans le pays et va l'être de plus en plus au moment où le pays s'apprête à rembourser. Parce que oui, il faut rembourser. Et il faut le faire alors même que l'augmentation non maîtrisée des dépenses en sortie de Covid et de guerre en Ukraine a accentué considérablement pour la France les taux d'intérêt. Au final, entre 2022 et 2030, la charge de la dette va quasi doubler, atteignant plus d'un cinquième des recettes de l'État, c'est-à-dire 20% des recettes. Nous avons besoin d'argent. Il faut donc ouvrir un débat transparent, de manière pragmatique sur les recettes. Or, le PSMT n'a rien documenté sérieusement. Je pense par exemple au fait que le Trésor a commis il y a quelques années une étude sur la TICPE, l'assise sur l'énergie, dont nous savons que son rendement va baisser d'un tiers entre 2022 et 2030. Par quoi cet argent en moins va-t-il être compensé ? Rien n'est défini. En supprimant les niches fiscales sur le gazoil professionnel, le gazoil agricole par exemple, ou en augmentant la TVA comme certains le suggèrent. Nous ne le savons pas. Pire, Cette absence de débat et ce refus des réformes structurelles sur la fiscalité coïncident avec les problèmes de calculettes de Bercy. Cela a été évoqué par mes précédents orateurs. Cela fait trois ans maintenant que nous vivons les mêmes séquences, celles d'un budget erroné nécessitant des arbitrages en catimini, quelques semaines seulement après les débats démocratiques du pays. Parce que votre politique en définitive est claire. c'est celle de renvoyer les arbitrages budgétaires sur le seul volet dépenses. Or, de ce point de vue, si nous avons des désaccords, et c'est normal en démocratie, nous pourrions nous attendre au moins à voir des débats de réformes structurelles à minima, celles qui sont inscrites dans le PSMT. Mais non, il y a dans le PSMT un certain nombre d'axes de réforme, mais nous ne voyons toujours rien venir à l'agenda du Parlement. Aussi, alors que le budget de 2026 s'annonce comme la quadrature du cercle. Depuis janvier, telle sœur Anne, nous ne voyons toujours rien venir. Au contraire, le gouvernement appuie des deux pieds à fond sur la pédale du statut quo. On a une réduction des séances de travail parlementaires au strict minimum. On a des textes sur les processus électoraux ou sur la sécurité, mais nous ne voyons rien en termes de réorganisation du pays. Et là encore, d'un côté, si nous ne voyons rien, ce qui est vrai, c'est que tous les jours, quand nous allumons le poste, médiatiquement, nous voyons ici une sonde jetée en l'air, où là, une nouvelle idée de modification structurelle. Mais dans les faits, aucune annonce, aucun texte, aucun projet. Dit autrement, pour faire Une analogie avec l'alpinisme, nous sommes face à l'Himalaya et d'un côté on refuse à l'alpiniste tout apport nutritionnel supplémentaire mais de l'autre vous lui maintenez toute la charge. C'est curieux comme mode de gestion parce que nous savons dès à présent que ça ne passera pas. Ça pose donc un problème de sincérité budgétaire. Alors de facto, À quoi assistons-nous ? À la technique du rabot. On rabote les niches fiscales, on rabote les dépenses. Et c'est là le plus terrible. D'une part parce qu'en rabotant, vous allez au plus facile. C'est-à-dire que ce sont les budgets d'investissement qui sont dans la cible. On le voit, France 2030, transition écologique, recherche et enseignement supérieur, aide au développement. Voilà la façon dont vous préparez l'avenir. Supprimer les dépenses d'investissement. en rabotant budget après budget tout ce qui nous aiderait pourtant donc à surmonter les défis de demain. Mais pire, et je termine mon propos, parce que d'autre part vous empêchez la France d'être au rendez-vous de son défi budgétaire, la procrastination aboutit à renvoyer aux autres. les arbitrages forcément plus douloureux demain. Est-ce que c'est cela la responsabilité ? Nous ne le croyons pas. Non seulement avec ce mode de gestion de non-choix, vous ne parvenez pas à boucler le budget, mais en plus, vous créez les conditions de l'instabilité politique. C'est le principal problème à nos yeux. Merci. La parole est maintenant Madame Florence Blatrix-Contat pour le groupe socialiste écologiste et républicain. Vous avez neuf minutes, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le groupe socialiste, écologiste et républicain aborde l'examen de ce rapport d'avancement annuel du PSMT 2025-2029 avec une double exigence, d'une part la lucidité face au déséquilibre budgétaire, d'autre part la conviction que des choix budgétaires doivent impérativement servir la justice sociale et et la transition écologique. Car derrière les chiffres du déficit, ce sont des enjeux concrets qui se jouent, la qualité de nos services publics, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français et notre capacité collective à relever les grands défis du siècle. Le constat d'abord, les chiffres sont sévères. un déficit de 5,8% du PIB en 2024, bien au-delà des prévisions, une dette publique qui dépasse allègrement les 110% du PIB, des prévisions de croissance systématiquement revues à la baisse. La Cour des comptes parle d'une dérive inédite et d'une année noire pour 2024. forçait de constater que cette perte de contrôle budgétaire illustre une forme d'improvisation permanente incompatible avec la nécessité d'une stratégie claire et de long terme. Face à ce constat alarmant, le gouvernement nous présente aujourd'hui une trajectoire corrigée pour les années à venir. Désormais, l'objectif est donc de ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026, en 2026, puis progressivement 4,1% en 2027, 3,4% en 2028, et de conserver le cap des 2,8% en 2029. Inutile de rappeler que cette trajectoire s'écarte largement de la loi de programmation des finances publiques, aujourd'hui très largement obsolète. En ce qui concerne la charge de la dette, elle est estimée à 53 milliards en 2025, mais sa trajectoire reste incertaine. La volatilité des taux d'intérêt nourris par des incertitudes internationales ouvre un champ des possibles instables et potentiellement dangereux. Dans ces conditions, l'inversion du ratio dette sur PIB annoncé pour 2028 nous paraît là encore très aléatoire. S'agissant des hypothèses de croissance, reconnaissons qu'elles sont plus réalistes que celles des précédents gouvernements qui frôlaient l'aveuglement avant de se heurter au mur de la réalité. Le gouvernement table désormais sur 0,7% pour 2025, puis entre 1,2 et 1,4 les années suivantes. C'est, selon le Haut Conseil des finances publiques, légèrement supérieur au consensus des économistes, mais c'est déjà une première leçon tirée des erreurs passées. Personnellement, je regrette toutefois que le gouvernement table à nouveau sur une fourchette plutôt haute, malgré l'accumulation des risques, car il faut rester lucide. ni la conjoncture internationale, ni le le poids croissant du dérèglement climatique sur notre économie, ni les tendances démographiques actuelles ne justifient un optimisme excessif dans le quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive, la prudence devrait rester de mise car si nous savons toujours quoi faire des bonnes surprises, nous avons beaucoup plus de difficultés à gérer les mauvaises surprises. Sur les économies annoncées 40 milliards d'ici 2026, le flou reste important. Les mesures concrètes font cruellement défaut et les tableaux de suivi restent désespérément vides. En réalité, nous sommes invités à débattre d'une trajectoire dont les fondements restent à bâtir. Pire encore, les rares mesures identifiées frappent toujours les mêmes, réformes de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, des retraites, autant de recul sociaux que le gouvernement, avec cynisme, préfère présenter sous le label « soutien à l'emploi ». Aucun chiffrage précis des économies attendues n'est d'ailleurs avancé, ce qui nuit gravement à la transparence de ce rapport d'avancement et empêche toute évaluation sérieuse de la trajectoire présentée. Plus fondamentalement, le gouvernement ne prend pas la mesure de la gravité de la crise budgétaire qu'il a lui-même provoqué. Ils persistent à écarter toute réponse sérieuse qu'il s'agisse de remettre en cause les dépenses fiscales inefficaces ou de faire davantage contribuer les grandes entreprises et les ultrariches sur le modèle de la taxe Zuckman. Une fois encore, le gouvernement préfère reporter l'effort sur celles et ceux qui sont déjà durement touchés par les reculs sociaux. Ce document est une démonstration supplémentaire de la poursuite de la politique conduite depuis sept ans. Un INI qui se veut équilibrer mais qui, en réalité, défend les intérêts des plus puissants tout en exigeant toujours plus de ceux qui supportent déjà l'essentiel du fardeau. La question du partage de l'effort budgétaire entre les ménages et les entreprises reste également en suspens. L'évolution du taux de prélèvement obligatoire, avec une hausse sur les revenus des ménages et une stagnation pour les entreprises, soulève de sérieuses interrogations quant à l'équité de notre système fiscal et à son efficacité pour soutenir la demande intérieure, moteur pourtant essentiel de la croissance. Plus généralement, il est permis de douter de l'efficacité d'une politique de l'offre qui, malgré un endettement record, ne semble pas avoir restauré la confiance des investisseurs dans notre économie. Nous pouvons également regretter l'absence de détails concernant les niches fiscales visées par le gouvernement. Par ailleurs, le rapport d'amancement consacre plusieurs pages à une analyse par sous-sector des administrations publiques. On y lit que les collectivités territoriales seraient responsables d'une large part du dérapage. C'est une lecture partielle, voire erronée. En réalité, nous le savons, cette situation résulte principalement de l'accélération des investissements locaux liés au cycle électoral. C'est un cycle récurrents récurrents et c'est nécessaire. Ces dépenses ne sont pas des dérives mais bien des investissements d'avenir, des équipements publics, équipements pour la transition énergétique, pour les services de proximité. Les collectivités jouent un rôle essentiel d'aménageurs du territoire et de remparts sociaux. Alors je le dis clairement, il est temps d'arrêter d'opposer l'État et les collectivités. Madame la Ministre, le redressement durable des comptes passera par une mobilisation conjointe et un respect de l'autonomie locale. Je voudrais enfin consacrer la dernière partie de mon intervention à une question essentielle, celle des marges de manœuvre dont l'État doit impérativement disposer pour réussir la transition écologique et la réindustrialisation du pays. Or, il est pour le moins préoccupant de constater que la priorité affichée à la réindustrialisation peine à se traduire dans les actes. L'annonce récente par ArcelorMittal de la suppression de centaines de postes en France en est une illustration éclatante juste après l'abandon de Vancorex. C'est la poursuite d'une désindustrialisation que nous voyons. Donc, on a une véritable fragilité de notre appareil productif qui traduit un manque d'ambition en matière d'investissement. De même, concernant la transition écologique, aucune indication n'est donnée sur une trajectoire d'investissement à réaliser dans les années à venir. Pourtant, il existe une dette irréversible, c'est bien la dette écologique. Madame la Ministre, chaque investissement retardé, chaque engagement repoussé, nous rapproche inexorablement. En conclusion, En conclusion, j'ajouterai que ce rapport d'avancement révèle l'échec d'une politique budgétaire qui accumule des paradoxes. Elle creuse la dette sans relancer l'investissement. Elle aggrave les inégalités sans redresser les comptes. L'analyse du groupe socialiste écologiste et républicain est sans appel. Cette spirale négative ne sera brisée que par un changement de cap. Le nécessaire redressement de nos finances publiques ne peut se faire au détriment des investissements. Nous devons oser investir massivement dans notre appareil productif, notre formation professionnelle, notre défense, mais également dans les transitions écologiques et numériques, car c'est précisément cette absence d'investissement qui condamne notre économie à la stagnation et nos finances publiques au déficit chronique. Cette relance exige une réforme fiscale courageuse, mettant fin aux rentes qui privent l'état de ressources nécessaires. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Marc Lamini pour le groupe Les Indépendants, République et territoires. Vous avez six minutes, cher collègue. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général du budget, madame le rapporteur général de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. Le rapport d'avancement annuel sur le plan budgétaire et structurel de moyen terme pour les années 2025 à 2029 est un document technique. Nous l'avons examiné ce matin en commission des finances et le titre, et je salue bien sûr le travail du rapporteur général et de l'ensemble des services de la commission, intitulé un déficit public trop élevé mais une trajectoire de dépenses nette tenue. C'est un dossier que le gouvernement soumet à Bruxelles pour montrer à nos institutions européennes que même si nous ne respectons pas les règles budgétaires que nous avons fixées en commun, nous faisons preuve de bonne volonté et d'action. Ces règles budgétaires européennes, nous les connaissons ici tous. Le déficit public annuel ne doit pas dépasser les 3%, tandis que la dette publique doit, quant à elle, restait inférieure à 60% du PIB. En 2024, notre déficit fut de 5,8% et notre dette représentait 113% de notre PIB. C'est dire si le chemin à parcourir est long. Mes chers collègues, respecter ces engagements auxquels nous sommes soumis nous paraît aujourd'hui être un rêve inatteignable, tel le mythe de Sisyphe. qui ne parvient jamais à rouler son rocher jusqu'en haut de la montagne. Pourtant, si l'on coparde notre déficit et notre dette avec nos amis européens qui sont soumis aux mêmes règles que nous, on constate immédiatement qu'une grande partie d'entre eux parvient à respecter ces engagements budgétaires. Pour ne prendre que cet exemple, 16 des 27 pays de l'Union européenne ont en 2023 des déficits inférieurs à 3% du PIB, mais encore 4 pays ont affiché un excédent Rappelons-nous, mes chers collègues, de la crise financière de 2008, puis de la crise des dettes souveraines européennes. À l'époque, des détracteurs anglo-saxons avaient accusé quelques pays européens d'être en grande partie responsables de la crise européenne par leur manque de sérieux budgétaire. Il s'agissait du Portugal, de l'Italie, de l'Irlande, de la Grèce et de l'Espagne à l'époque. Les commentateurs mal intentionnés les appelaient les PICS. Laissez-moi donc vous parler, près de 20 ans après, de la situation budgétaire de ces pays. Le Portugal a été en 2024 en excédent budgétaire pour la deuxième année consécutive et les analystes projettent une année 2025 qui finira elle aussi en excédent budgétaire. L'Irlande a eu un excédent de 23 milliards d'euros, soit 4,7% de son PIB en 2024 après une année 2023 où elle a déjà dégagé 10 milliards d'euros Comme la France, l'Italie ne respecte pas les traités mais elle peut s'appuyer sur une balance commerciale que nous lui envions. Finissons par la Grèce et l'Espagne. Après des années particulièrement compliquées, ces deux pays respectent désormais les traités en ayant des déficits inférieurs à 3%. qu'ont fait ces pays pour changer la donne. Rien que nous ne puissions faire, réformes économiques, allègements du poids de l'étoile et baisses des prélèvements pesant sur le tissu entrepreneurial. Mes chers collègues, il n'y a aucune fatalité dans la gestion budgétaire. Qui est le mauvais élève aujourd'hui peut montrer le bon exemple demain. Nous avons donc étudié avec attention ce rapport d'avancement annuel sur le plan budgétaire et structurel de moyen terme du pays. Il nous apprend beaucoup de choses. Nous y apprenons que le gouvernement engagé cet automne avec l'aide des sénateurs des mesures de redressement à hauteur de 50 milliards afin de ramener le déficit à 5,4% en 2025 après une année 2024 où nous avons connu un déficit à 5,8%. La nécessaire baisse de nos dépenses publiques est désormais une évidence pour tout le monde et les Français nous soutiennent. Les économies engagées en 2025 sont un bon début mais il ne faudrait pas s'arrêter là. La marche est dure et sera longue mes chers collègues. mais il nous faut avancer pas à pas sans jamais faire demi-tour. C'est pour ça que vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, c'est à ce prix aussi que nous pourrons nous aussi, à notre tour, rentrer dans les clous d'une bonne gestion budgétaire et respecter nos engagements envers nos partenaires européens. Enfin, et j'en finirai par là, Baisser nos dépenses de fonctionnement en particulier, vous l'avez rappelé Madame la Ministre, de budget fondamentaux, budget de la sécurité sociale, budget de l'État. Baisser nos dépenses, c'est bien plus que respecter des engagements budgétaires, c'est redonner des marges de manoeuvre à notre pays pour agir là où c'est nécessaire quand ça l'est, par exemple, pour rembourser une dette qui atteint 113% de notre PIB et pour des mesures de financement essentielles, l'éducation nationale, le réarmement, la sécurité, la santé ou notre transition écologique, sans oublier aussi le soutien en direction des collectivités territoriales au temps de missions fondamentales indispensables. Voilà donc c'était un petit peu le point de vue de notre groupe des indépendants et je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Stéphane Sautarelle pour le groupe Les Républicains. Vous avez six minutes, chers collègues.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame, Monsieur, les rapporteurs. La réforme du pacte de stabilité et de croissance prévoit la réalisation par les États membres d'un plan budgétaire et structurel à moyen terme pour la période 2025-2029. Le respect de la trajectoire prévu par ce dernier suppose la production d'un rapport d'avancement annuel, objet de notre débat du jour, publié en 2025 pour la première fois et qui détaille les prévisions financières et les réformes envisagées pour garantir le respect de la trajectoire globale du PSMT. Étant concerné par une procédure de déficit excessif, la France doit veiller au respect de la trajectoire définie dans son PSMT. La réduction du déficit public de 5,8% entre 2024 et 5,4% en 2025, permet à la France de garantir le respect de la trajectoire du PSMT, mais sur une nouvelle échelle. Surtout, la trajectoire présentée jusqu'en 2029, nous devons prendre acte, permet de respecter le critère d'évolution de la dépense publique sur les dépenses suivantes. On en est seul, comme en cumul d'exercices. Pourtant, la situation de la France reste bien préoccupante et bien loin de la loi de programmation pluriannuelle. suppose désormais un effort d'ajustement des finances publiques de 110 milliards d'euros à l'horizon 2029 contre seulement 50 milliards en 2022. Le dérapage du déficit public en 2023 et en 2024 en est noir s'il en est, a un effet conduit à plus que doubler l'effort d'ajustement nécessaire pour amener le déficit sous les 3%. Principal inquiétude, la dette. Le ratio d'endettement dépasse 125 % du PIB en 2029 et s'approcherait du seuil de 130 points du PIB dès 2031. En particulier, la charge de la dette augmenterait continuement pour atteindre 3,4 % du PIB en 2029, soit 112 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des budgets cumulés d'éducation nationale et de la défense. Il est donc nécessaire de respecter la trajectoire actuelle et d'engager l'effort de redressement de 110 milliards d'euros d'ici à 2029, en ce que tout retard supplémentaire rendra les ajustements indispensables encore plus importants et difficiles. L'année 2025 est donc déterminante pour enfin amorcer une trajectoire sérieuse de redressement des finances publiques après deux faux départs en 2023 et en 2024, avant que nous ne subissions une austérité imposée si nous ne parviennions pas à trouver des solutions par nous-mêmes. Il est un effet urgent de restaurer la crédibilité des engagements de la France en matière de finances publiques, pour éviter une hausse incontrôlée de la charge de la dette qui atteint déjà près de 59 milliards et qui augmente et qui augmente sous l'effet de son propre poids et résorber par ailleurs la divergence avec nos partenaires européens. Cela a été dit, la France reste hélas. en effet le cancre de l'Europe. Alors que l'année 2025 doit être celle de la préparation de réformes de structure et d'un budget ambitieux pour 2026 afin de garantir le respect de la trajectoire du PSMT, les réformes présentées par le gouvernement apparaissent insuffisantes et bien limitées. Les efforts budgétaires pour 2025 ne sauraient être reconductibles. La hausse des prélèvements obligatoires tels qu'opérés reposent principalement sur des mesures temporaires, parfois circonscrites au seul exercice 2025, et pèsent fortement sur les contribuables. Quant aux réductions de dépenses réalisées, elles s'appuient majoritairement sur des coûts de rabots dont la reconduction pour les prochains exercices n'est ni garantie et surtout ni souhaitable, et qui les impactent sans en renforcer l'efficience et surtout sans cibler les crédits improductifs. Cela nécessite de penser la question de la répartition des efforts, l'assainissement des finances publiques ne pouvant peser sur le potentiel de croissance à moyen terme via des hausses de prélèvements obligatoires disproportionnés ou des réductions de dépenses défavorables à l'activité économique. Les réformes proposées par le gouvernement en gage de crédibilisation du respect de la trajectoire du PSMT dans le rapport apparaissent trop insuffisamment documentées et peu à même de garantir une consolidation à hauteur de 110 milliards d'euros. La volonté politique semble encore, hélas, bien absente dans un océan d'incertitude qui nous submerge, certes, mais qui montre surtout une impuissance coupable et que nos concitoyens ne comprennent plus. Vous vous contentez à l'effet de proposer pour 2026 une nouvelle méthode de réalisation de revues de dépenses et un examen plus approfondi des niches fiscales. Certes, toutefois, ces exercices ont déjà été menés au cours des années récentes avec des résultats en 2010. Sans choix politique clair et ambitieux, ces propositions ne sauraient être significatives à l'échelle budgétaire. De même, les propositions de réforme que vous présentez dans le rapport apparaissent très vagues, sans chiffrage, ni études d'impact financier et peu à même de crédibiliser la démarche budgétaire générale. L'urgence est donc aux réformes structurelles, particulièrement en matière de régulation des dépenses sociales, qui pèsent plus qu'ailleurs en Europe sur nos finances publiques. et de refondre des relations financières entre l'État et les collectivités, mais cette fois, sans les spolier, tant la dépense locale reste la seule garante de services publics et d'investissements pour l'avenir. L'absence des vocations d'une réelle réforme de l'État et de notre système social au sein du rapport interroge sur votre volonté politique comme sur votre capacité à respecter la trajectoire nécessaire via PSMT. Faire des choix ou subir, voilà ce à quoi nous sommes confrontés collectivement et nous souhaitons y répondre avec justice et courage. Ces débats, j'en termine par là, nous épuisent, épuisent nos concitoyens et je crois qu'aujourd'hui, l'heure des choix est arrivée et non plus du partage de la pédagogie qui, je pense, est bien perçue par chacun. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Stéphane Foissin pour le Groupe RDPI. Vous avez six minutes, cher collègue.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure générale, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Le rapport d'avancement sur notre trajectoire budgétaire confirme l'engagement déterminé du gouvernement pour restaurer nos finances publiques, malgré un contexte économique international incertain. Après avoir atteint 5,8% du PIB en 2024, le déficit est en voie d'être réduit à 5,4% cette année grâce à un effort majeur de maîtrise des dépenses de l'État et des collectivités. En moyen terme, l'objectif est clair, ramener le déficit public à 4,6% en 2026, puis sous la barre des 3% d'ici 2029 conformément aux ambitions du plan budgétaire et structurel. La trajectoire présentée dans ce rapport permet de respecter l'évolution de la dépense primaire nette recommandée par le Conseil européen, engagement crucial jusqu'en 2029. Je tiens d'ailleurs à saluer la rigueur du gouvernement qui parvient à maintenir la croissance de cette dépense à 0,9 et ce malgré les incertitudes économiques mondiales, hausse des droits de douane, tension internationale et financière, si le déficit n'est pas encore une espèce protégée et l'est désormais traité avec prudence et méthode. Cependant, nous devons veiller à ce que cet effort collectif bénéficie à tous nos territoires. Le souci d'équité territoriale doit continuer à guider notre action. Les ajustements nécessaires ne doivent pas aggraver les fragilités existantes, notamment dans les territoires ultramarins et ruraux, qui connaissent des réalités économiques et sociales particulières. Le gouvernement a déjà montré sa vigilance sur ce point, mais nous devons poursuivre et amplifier cette dynamique. A ce titre, je salue les efforts déjà réalisés pour associer les territoires à la mise en œuvre des politiques publiques et je forme le vœu que cette démarche de co-construction soit amplifiée. La réussite du redressement passe par l'adaptation permanente aux réalités locales, par l'écoute de nos élus de terrain et par l'accompagnement différencier de nos concitoyens. En tant que médecin, je suis particulièrement attentif aux réformes entreprises dans notre système de santé. Les mesures contre les déserts médicaux, la lutte contre la pénurie de soignants et les investissements dans les établissements médicaux sociaux sont absolument essentiels. Usages renforcés de l'intelligence artificielle pour améliorer la pertinence des prescriptions ou encore le suivi des patients d'infection longue durée sans médecin traitant vont dans le bon sens. Mais veillons à ce que ces réformes soient concrètes et adaptées aux réalités locales, car un système de santé et performance est d'abord un système proche, humain et réactif partout sur le territoire. De la même manière, la prise en compte des spécificités locales dans les politiques de transition écologique, notamment pour les territoires ultramarins, illustre une approche pragmatique et juste de la transformation de notre modèle économique. Il s'agit de construire une écologie de solution respectueuse des contraintes et des atouts de chaque territoire. Il conviendra néanmoins de renforcer cette logique dans les politiques de soutien à l'emploi. Dans les territoires où le chômage structurel reste élevé, des dispositifs adaptés doivent continuer à être développés pour éviter tout effet d'éviction et garantir que l'effort national en faveur de l'emploi bénéficie pleinement aux plus fragiles. Le travail doit demeurer un puissant levier d'émancipation et de cohésion sociale. J'invite donc le gouvernement à prolonger avec la même exigence et la même ouverture l'association des territoires à l'évaluation et à l'ajustement de ces politiques publiques. Car les succès de demain s'écriront dans la co-construction et dans l'adaptation permanente aux réalités de terrain. Le groupe RDPI apporte donc son plein soutien à ces trajectoires responsables et ambitieuses et continuera d'être un partenaire exigeant et engagé pour en assurer le succès aux services de tous les Français. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Raphaël Dobé pour le groupe RDSSE. Vous avez cinq minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs généraux, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Ce rapport sur la trajectoire de nos finances publiques dresse un état des lieux sans complaisance, et tant mieux. Tant mieux parce que la lucidité est évidemment le premier pas sur le chemin de la solution. Alors oui, les défis auxquels notre pays doit faire face sont immenses, et vous le savez, mais la lucidité ne suffit pas, et nous attendons désormais une volonté politique. Sortir la France de la stagnation économique et du surendettement, oui, c'est impératif, Mais sortir aussi les Français de cette espèce de désespérance financière et de l'anxiété qui nous plombe au quotidien, voilà ce qu'on attend de la volonté politique. La seule voie de l'austérité, celle du serrage de vices budgétaires, celle des mauvaises nouvelles et des horizons tristes, ne peut pas suffire. Donc mon groupe partage l'objectif d'assainissement de nos finances publiques, mais nous refusons tout fatalisme budgétaire qui s'appuierait sur des projections technocratiques pour figer notre action. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que les projections sont bourrées d'incertitudes. On l'a vu avec les estimations de recettes de l'exercice 2024. Aujourd'hui, l'environnement international aggrave considérablement le risque d'erreur. Mais il y a 6 mois déjà, je m'inquiétais à cette tribune des hypothèses de croissance au regard des remontées du terrain et de 1,1%. On est aujourd'hui à 0,7%. L'exécutif est tenu par ses prévisions de croissance et fait le choix du repli, par crainte légitime de sortir des clous budgétaires, comme on vient de le voir avec l'annulation de plus de 3 milliards d'euros par décret. Cela concerne des missions aussi essentielles que la recherche, l'économie, l'agriculture ou, comme toujours, l'aide au développement. Cette navigation à vue, toujours moins disante, produit des économies non pérennes, sans stratégie d'ensemble et nous prive des réformes structurelles nécessaires. Alors il est vrai qu'on annonce 3 milliards d'économies par la suppression ou la fusion d'un tiers des agences de l'État. Le groupe RDSE se réjouit d'avoir eu raison trop tôt lorsque Jacques Mézard publié son rapport sur les autorités administratives indépendantes il y a 10 ans. Mais là encore, il nous semble que la prudence est de rigueur dans les économies attendues. La deuxième raison pour laquelle nous refusons le fatalisme budgétaire, c'est qu'il en appelle aux efforts de tous, mais qu'il ne se traduit pas toujours en mesure de justice fiscale. On vient de le voir avec l'exemple édifiant de la taxation des dividendes, où Bercy contourne allègrement la volonté du législateur pour laisser perdurer une pratique frauduleuse. Le redressement de nos comptes publics ne peut pas renoncer au levier des recettes, ni à répondre à la demande de justice fiscale qu'implore la classe moyenne française. La situation budgétaire est directement liée à des baisses de fiscalité. Il n'y a pas d'autre solution que de revenir en partie dessus. Enfin, nous refusons le fatalisme budgétaire parce que la méthode du rabot qui l'accompagne présente un risque récessif pour l'économie et ne prépare absolument pas l'avenir. Financer la mutation énergétique et industrielle, investir dans l'innovation et la recherche pour retrouver de la compétitivité, assurer notre sécurité. Au fond, ce que dit ce rapport est aussi instructif que ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas comment mobiliser le levier des recettes, pourtant indispensable à la préservation de notre modèle social républicain, qui exige évidemment davantage d'efficience, mais dont la force est indiscutable, de même que l'attachement que voulent les Français. Ce modèle a un coût qu'il nous faut assumer collectivement. Ce rapport ne dit pas comment la France va garder demain une capacité de réaction et d'ambition. Or, c'est toute la question. Se contenter de gérer la pénurie prépare le déclin. Prenons exemple sur certains de nos voisins européens. Ce rapport ne dit pas ce que sont les réformes structurelles qui, seules, peuvent rendre à partir de 2030 la dette soutenable. La charge de la dette va augmenter jusqu'en 2028. Sa soutenabilité repose sur l'hypothèse que le plateau historiquement haut où elle se trouve sera suivi d'une décrue prolongée au-delà de 2030 pendant au moins dix ans. Je le dis très tranquillement, cette décrue n'aura pas lieu sans réforme profonde dans les trois ans qui viennent. Voilà en quelques mots ce que nous inspire la lecture de ce rapport. Réformons, travaillons, investissons. L'avenir nous appartient. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Michel Cannevet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez quatre minutes, chers collègues. Bien, monsieur le Président, madame et monsieur les ministres, chers collègues, Nous connaissons le paradoxe d'examiner un rapport annuel d'avancement des comptes publics alors même que ce document a été préparé il y a six mois seulement et alors même que la Commission européenne ne l'a valédée qu'il y a que trois mois. Mais c'est vrai que parmi les membres du groupe de l'Union Centrise, nous sommes particulièrement préoccupés par la situation des finances publiques, force est de constater que nous sommes échaudés par la situation que l'on a connue en 2024, l'année passée, au niveau des comptes publics. Je la rappelle, le vote en 2023 d'une loi de finances initiale, où on prévoyait un déficit à moins 4,4% du PIB pour arriver, vous le savez tous, à une situation à moins 5,8 %. Ceci appelle effectivement à ce que nous soyons en situation de vigilance extrême et c'est sans doute ce qui explique que nous soyons à ce moment précis en train de débattre de la situation financière des comptes publics dans notre pays. Alors c'est vrai, la situation est préoccupante. Le déficit qui est annoncé n'est pas dans les épures qui avaient pu être élaborées lorsque nous évoquions le plan à la loi de financement prévisionnelle des finances publiques 2023-2027. Je vous rappelle qu'il était prévu moins 3,7 pour 2025. Et même dans la version initiale du plan de stabilité de plan budgétaire et structurel à moyen terme, nous étions à un autre niveau que celui à partir duquel nous démarrons cette année. l'enjeu qui est devant nous pour faire en sorte que nous puissions apporter des réponses appropriées. Monsieur et Madame les Ministres, les défis devant nous sont extrêmement importants. Il y a la question de la transition écologique qui est absolument impérative et que nous appelons de nos voeux. Il y a la nécessité d'assurer notre sécurité, ce qui demandera des moyens. cela a été dit par les orateurs avant moi, la situation particulièrement préoccupante de l'ordonnement public. Le premier président de la Cour des Comptes nous le rappelait ce matin, 2 603 milliards de dette de l'État dont une partie va être à renégocier dans les années qui viennent avec sans doute un impact extrêmement significatif sur notre capacité à agir demain pour pouvoir mener des politiques publiques qui sont nécessaires comme je viens de l'évoquer. Et c'est donc un effort qui demandera du courage, madame et messieurs les ministres, pour justement faire en sorte que nous arrivions à réduire la dépense publique dont tout le monde dit qu'elle est particulièrement élevée. En tout cas, les statistiques en regard des autres pays autour de nous le montrent bien. Le journal Les Échos, il y a trois jours, nous donnait le bonnet d'âne des pays de la zone euro, faut-il le rappeler, c'est dire l'effort et le courage qu'il faudra avoir pour proposer des réformes structurelles qui seraient nécessaires, mais dont le contexte politique n'est sans doute pas le plus favorable. Mais il va falloir agir en ce sens. Et vous pouvez compter sur les membres du groupe de l'Union centrale pour assembler un certain nombre de propositions. Vincent Delahaye reviendra tout à l'heure. Et puis au plan économique, nous misons beaucoup, c'est vrai monsieur le rapporteur général, sur la nécessité de favoriser l'entreprenariat et l'activité économique dans notre pays. Celle-ci est clairement entravée par des contraintes administratives de taux de nature. Et une partie de la clé de réponse aux besoins financiers auxquels nous avons à faire face, parce que nous ne partageons pas l'idée qu'il faut augmenter les impôts, c'est qu'il y ait une croissance qui permette de générer des ressources. Et cela peut se faire parce que nous avons de la volonté dans notre pays, nous avons des acteurs qui sont prêts à y aller, mais nous avons des entraves administratives, il faut les lever. Merci de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est maintenant monsieur Pierre Barros pour le groupe CRCK. Vous avez cinq minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, chers collègues, nous débattons aujourd'hui du plan budgétaire et structurel de moyen terme et de son actualisation à travers le rapport d'avancement annuel adressé à notre Commission. Ces deux documents Nous n'en sommes pas là pour en remettre en cause leur technicité. Ici encore, c'est l'esprit ayant présidé à la conception de ce rapport qui nous préoccupe fortement. À chaque ligne, nous découvrons un renoncement de plus. C'est l'abandon de toute ambition économique, sociale et démocratique. Vous avez fait vos choix, les faits sont là. Depuis 2017, nous assistons à une baisse tendentielle des recettes publiques par la suppression de l'ISF, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le plafonnement de la fiscalité sur les dividendes. A cela s'ajoute un stock d'aide directe de niche fiscale et d'exonération sociale aux entreprises qui oscillent entre 180 et 250 milliards d'euros par an selon la cour des comptes. court des comptes qui confirment également qu'à la moitié du déficit public provient aussi bien de la baisse des prélèvements obligatoires. Nous sommes face à un continent budgétaire où se mêle l'injuste, l'inefficace et l'injustifiable. Et pourtant, vous ne revenez pas sur ces choix. Vous prétendez rétablir les comptes sans jamais toucher à ce gisement. Votre choix, ce n'est pas celui d'une politique d'équilibre, votre choix, c'est celui d'une politique de classe. L'ajustement budgétaire que vous projetez atteint 110 milliards d'euros d'ici 2029. En 2026, il faudra trouver 40 milliards. Vous les chercherez, une fois encore, dans les services publics, dans les dépenses sociales et au détriment des collectivités. C'est ainsi que vous avez annoncé le week-end dernier, sans prendre le soin d'en débattre réellement avec le Parlement, l'annulation de 3,1 milliards d'euros de crédit qui a été alloué aux collectivités. Les aides à l'investissement, tel le fond vert, la politique de la ville, sont les plus impactées. Et que dire de la suppression des politiques publiques et la fusion des agences de l'État que vous annoncez dans la presse pour fin décembre 2025. Le tout sans toucher ni aux rentes, ni au super-profit. Sans regarder du côté de l'organisation de notre administration centrale et déconcentrée, ce n'est pas l'État qui ajuste ou qui s'ajuste, c'est la société qui trinque. Le capital, lui, reste intouché, intouchable. Les vérités, c'est que la dette est brandie comme une menace permanente pour imposer l'austérité comme seul horizon, alors qu'elle devrait engager une réflexion collective et structurelle sur l'investissement, mais aussi sur le fonctionnement. C'est un principe pour les Français. On leur explique que les caisses de l'État sont vides, que les Françaises et les Français doivent travailler plus, doivent faire des efforts, et ensuite ils découvrent stupéfait, la clause de sauvegarde pour financer l'effort militaire. Alors, chers collègues, une question meute à rôde. Pourquoi cette clause ne pourrait-elle pas être activée pour la bifurcation écologique, pour la réindustrialisation, pour la justice sociale ? Ces sujets ne sont-ils pas tous essentiels pour notre avenir et celui de nos enfants ? Car enfin, et en effet l'histoire, notre histoire, nous a enseigné qu'un pays ne tient pas durablement sur le déséquilibre de ses efforts. Dans un contexte économique des plus difficiles et des plus inédits pour la plupart des Français, vous annoncez de nouvelles coupes pour l'éducation, le logement social, les mobilités du quotidien, tout en envisageant une hausse de la TVA, un gel du point d'indice ou encore un affaiblissement de la solidarité locale. Coupé dans la santé, coupé dans les retraites, c'est transférer des dépenses socialisées vers des dépenses privées et cela remet en cause profondément notre modèle social de couverture universelle pour toutes et tous. Tout cela est-il bien sérieux ? Tout cela est-il bien raisonnable ? Tout cela est-il bien responsable ? Ou jeter de l'huile sur un brasier social déjà incandescent en créant la pénurie ? Pénurie d'enseignants, pénurie de logements, pénurie de soins, pénurie de temps et de sens pour les agents publics. Dans le même temps, vous confortez les dividendes. Le patrimoine des plus grandes fortunes est multiplié par 5 depuis 2009 et 100 milliards d'euros sont distribués aux actionnaires du 440 en 2024. C'est la fracture de la France que vous organisez. Vous ne faites d'ailleurs pas que l'organiser, vous la confortez. Vous confortez cette fracture sociale en faisant fi chaque année de la vie des Français par le refus d'un vote démocratique de votre budget au Parlement. Chers collègues, une autre voie existe évidemment, celle de la réorientation budgétaire fondée sur la justice fiscale, celle d'un état stratège qui se préoccupe davantage des conditions de mise en œuvre des politiques publiques, celle de l'investissement massif dans la transition écologique, dans la santé, dans les savoirs. Celle de la coopération industrielle dans une logique de partage technologique et de bifurcation productive. En bref, nous avons besoin d'une politique du futur, là où vous persistez à administrer le passé. Nous ne souffrirons donc pas à ce plan, nous ne l'amenderons pas, nous le refusons dans son principe, dans ses méthodes et dans ses conséquences. Je vous remercie. Merci, Merci, cher collègue. La parole est maintenant à madame Christine Lavarde pour le groupe des Républicains. Vous avez 7 minutes, cher collègue. Merci Monsieur le Président. Donc force est de constater que ce débat s'inscrit dans une dynamique positive quant au contrôle de la dépense publique. En effet, il concrétise la vision d'un Parlement davantage mobilisé sur l'analyse de l'exécution budgétaire, vision qui avait d'ailleurs guidé la révolution de la LoL en 2021, par la fusion du débat d'orientation budgétaire et du débat sur le programme de stabilité en une séquence unique aujourd'hui désormais consacrée à l'évaluation. Ce débat est le premier à s'attacher au contrôle du respect de la trajectoire de finances publiques présentée en octobre dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme, né de la né de la réforme du semestre européen. Et la pratique budgétaire elle-même évolue dans une bonne direction depuis quelques mois. Après deux exercices marqués par d'exceptionnels dérapages des comptes publics que je pense que notre Commission a largement documenté et une incapacité absolue à freiner l'évolution des dépenses du champ social ou à accompagner efficacement les collectivités face à leurs dépenses contraintes, le PLF et le PLFSS pour 2025 marquent un effort historique de près de 50 milliards. Cet effort, principalement porté par l'État, dont les dépenses devraient connaître en 2025 une quasi-stabilité en volume, mérite d'être souligné. à cet effort de consolidation et conjuguer la construction d'un nouveau cadre de pilotage des comptes publics qui associe enfin les parlementaires des commissions compétentes. Un comité d'alerte a été installé le 15 avril. Il faut poursuivre cet élan. En effet, la lecture de ce rapport d'avancement laisse poindre une crainte, celle que derrière ces évolutions rien n'est véritablement changé. L'heure n'est pas à l'autocongratulation. Je l'ai dit en février, le budget adopté pour 2025 était le pire à l'exception de tous les autres. Nous avons le devoir d'agir pour garantir la soutenabilité de la dette publique, pour renouer avec la crédibilité internationale qui trop souvent nous fait défaut, pour répondre aux immenses défis des transitions écologiques, numériques et démographiques. Alors cette exigence, elle nécessite d'atteindre la cible inscrite dans le PSMT, à savoir une consolidation de près de 110 milliards en 4 ans. Pour en assurer l'effectivité, sont égrainées une série de réformes pour les années à venir. Accélération de la transition écologique, modernisation de notre système de santé, renforcement de la lutte contre la faude, soutien de l'emploi, renforcement de la compétitivité. je suis obligée de constater que de PNR en PNR, de PNR en R2A, la documentation des réformes demeure lacunaire. Seule la sémantique utilisée évolue et encore à la marge. Ces éléments de langage satisferont peut-être les supervisaires européens, mais n'ont pas permis jusqu'à présent de rétablir nos comptes. Alors sans doute seront proposés, en soutien à ces orientations particulièrement peu précives, des stratégies ou des plans pluriannuels, des conventions ou des assises nationales de dialogue, des instances de suivi et de recommandation. s'y ajouteront aussi de nouvelles méthodes de réalisation de revues de dépenses. Alors là, non, il ne s'agit absolument pas d'une innovation majeure. Parce qu'entre 1946 et 2017, j'insiste sur 2017, le comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics s'est préoccupé de revues des dépenses. l'IGF a déjà réalisé des revues particulièrement pertinentes, dont on peut se demander si la seule utilisation n'est pas de caler les très nombreuses portes du navire amiral de Paul Chemetov. Alors là, tout cela n'est pas sérieux. Si nous pouvons nous satisfaire de l'effort consenti dans le budget 2025, la méthode employée pour en déterminer les modalités est à déplorer. Des coups de rabots, nos concertées, des choix, deux dernières minutes, le tout s'inscrivant dans le plus pur confort électoral. La consolidation d'ampleur qui nous attend, la défendance citoyenne ne peuvent nous laisser indifférents. Le temps n'est plus à la réformette paramétrique heureuse. Les dépenses sociales ne peuvent plus faire l'objet de simples mesurettes. Alors pourquoi ne pas refondre entièrement le système français de double couverture, tel que la Cour des comptes l'a formulé dans un rapport de juillet 2021, via la mise en place d'une restructuration du secteur des complémentaires santé et la création d'un bouclier sanitaire unique ? La sécurité sociale fait mieux que le secteur privé pour moins cher. Alors pourquoi persister dans un système de double cotisation et de double remboursement ayant prouvé son efficacité ? Les dépenses locales, elles ne peuvent plus être la variable d'ajustement de budget successif ni continuer de reposer sur un système devenu illisible, incompréhensible et inapte à favoriser des trajectoires d'investissement ambitieuses comme des efforts en fonctionnement. Fiscalité locale, dotation de l'État, mécanismes de péréquation n'ont pas besoin d'une énième conférence des parties prenantes ou vague de contractualisation. Elles appellent à une refonte complète. L'architecture de nos finances publiques, enfin, ne peut plus être conservée en l'État. Une consolidation aussi large que celle qui nous attend doit reposer sur un cadre financier, clair, lisible, intégré, pilotable. Les complexités effarantes du système actuel sont préjudiciables à l'objectif de ces atteintes. Par exemple, il est strictement impossible à la lecture des documents budgétaires d'établir un schéma des transferts de l'État aux collectivités ou à la sécurité sociale ou d'avoir une vue d'ensemble des comptes des administrations publiques tant d'un point de vue des recettes que des dépenses. Alors je vais vous donner un exemple, celui des collectivités. Pour recenser et retracer les 315 milliards de recettes des administrations publiques locales, il est nécessaire de réunir un total de sept documents que je vais vous lister. Le PSR figurant dans la première partie du PLF, les comptes de la mission RCT au sein de la deuxième partie et le compte de concours financiers avant ce collectivité. La fiscalité transférée et les taxes affectées qui sont elles sont recensées dans le tome 1 des voies et des moyens. Les dégrèvements et subventions qui eux sont disséminés au sein des missions ministérielles dédiées. Enfin les transferts entre ASSO et APULE qui eux sont inscrits au seul PLFSS, à l'instar du versement en mobilité. Et enfin toutes les recettes locales et subventions européennes dont le montant est uniquement précisé dans le rapport de l'OFGEL. dans le R2A, il est écrit que la trajectoire du PSMT sera respectée grâce aux réformes ultérieurement présentées par le gouvernement et adoptées par la représentation nationale. Mesdames la Ministre, Monsieur le Ministre, le Parlement n'est pas une simple chambre d'enregistrement. Il n'est pas admissible que le dispositif anti-coum-coum proposé par le rapporteur général, adopté à l'unanimité au Sénat et par la Commission mixte paritaire, soit à tellement détricoté par Bercy sous la pression de secteurs d'acteurs financiers. Alors en 1985 Jacques Delors avait osé innover avec les entretiens de Val Duchesse qui ont donné naissance au dialogue social européen. Alors force est de constater qu'à l'époque les organisations patronales étaient plutôt hostiles mais finalement elles ont accepté face à la mesure de la commission négocier ou nous légiférons. Alors aussi osant paraphraser Jacques Delors notre message est clair réformer avec audace réformer ou nous légiférons. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Vincent Delahaye pour le groupe de l'Union centrice. Vous avez quatre minutes, cher collègue.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame et Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, je vais vous dire des choses complémentaires à mon collègue Michel Canvet, dont je partage bien sûr le propos, mais je voudrais d'abord vous dire, Madame et Monsieur le Ministre, que votre volonté et votre souhait de redresser les finances publiques, c'est un discours que nous avons déjà entendu pas mal. Malheureusement, avec le bénéfice de l'âge, J'ai vu pas mal de ministres ici, sur ces bancs, nous dire à chaque fois qu'ils allaient redresser les finances publiques. Malheureusement, comme ce RAN, nous n'avons rien vu venir. Et au contraire, ça s'est plutôt dégradé. Et deuxième défaut un peu des discours que l'on entend sur les finances publiques, c'est toujours de dire que quand on regarde l'avenir, on reporte toujours les efforts un petit peu plus loin. Et je vais y venir un petit peu. Parce que à l'automne dernier, Le gouvernement Barnier nous a annoncé comme objectif d'être à 5% de déficit en 2025. Quand le gouvernement Bayrou est arrivé, on est passé à 5,4. Donc on n'avait plus qu'on a perdu 0,4. Et en réalité, comme les résultats ont été un petit peu meilleurs, même si c'est pas brillant du tout, pour 2024 on est à 5,8. En fait, l'effort en fait 0,4. Et qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? on est en train de nous dire qu'il va falloir faire le double, puisqu'il faudrait passer de 5-4 à 4-6, si je suis la trajectoire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on ne fait pas beaucoup d'efforts cette année, il va falloir en faire deux fois plus l'année prochaine. Moi je pense que c'est deux défauts qu'il faut absolument corriger. Alors, sur les dépenses publiques, puisqu'il faut s'attaquer prioritairement aux dépenses publiques, j'ai regardé les années sans crise. Parce que les années de crise, on a eu un flou artistique avec les dépenses exceptionnelles qui venaient se mêler aux dépenses ordinaires. J'ai regardé 2019. Avant crise, quel était le montant des dépenses publiques, monsieur le ministre ? 1348 milliards. 2024, quel est le montant des dépenses publiques ? 1670 milliards. Donc on a une augmentation de 322 milliards, je le dis pour mes collègues qui parlent d'austérité, en cinq ans, 322 milliards d'augmentation des dépenses publiques, ce qui fait 25% d'augmentation, si je sais calculer. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le ministre, on s'en était tenu à l'inflation, si nos dépenses publiques avaient évolué comme l'inflation, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Combien on aurait économisé ? Combien en 2024 on aurait économisé ? le bénéfice du calcul, c'est 120 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on serait à 120 milliards de moins si depuis 2019 nous avions fait évoluer nos dépenses en 2024 comme l'inflation. Je pense que c'est ça que nous devons tous avoir en tête. Parce que c'est très important, si on veut corriger l'évolution de nos dépenses publiques, il faut avoir ces éléments-là en tête. Et il y a deux choses qui me paraissent importantes en termes de dépenses publiques, et si nous voulons bien travailler avec vous, Madame et Monsieur le Ministre, c'est d'abord la transparence. La transparence, il faut qu'on soit informé. Le rapporteur général ce matin a dit qu'il y avait plus de transparence, je le note, mais ce n'est pas encore descendu aux membres de la Commission des Finances. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse avoir cette transparence. Ça veut dire que quand on dit qu'on gèle 8 milliards, on nous explique pourquoi 8 milliards et pourquoi pas 15, pourquoi pas 5. Quand on annule 5 milliards de réserves de précaution, ce qui n'est pas vraiment des économies, économies, pourquoi on fait 8 et 5 ? Ça fait 13. Pourquoi on arrive à 13 et pourquoi pas on arrive à 20 ? Et quand on dit 40 milliards pour l'année prochaine, comment sont calculés ces 40 milliards ? Moi j'aimerais bien avoir sur une feuille de calcul C'est 40 milliards. Et le dernier principe, j'ai pas le temps de le développer, j'avais que 4 minutes, mais c'est la prudence. La prudence dans les prévisions, mais on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres débats. En tout cas, je suis content d'avoir pu exprimer ici mon point de vue et le point de vue de l'Union centriste. Merci, cher collègue. Pour conclure le débat, la parole est à monsieur le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté nationale et du numérique. Monsieur Eric Lombard, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Sciences, Messieurs les rapporteurs généraux, je terminerai par là où vous avez terminé. Monsieur Delahaye, sur la prudence. Et effectivement, le rapporteur général, cher Jean-François Lisson, vous avez commencé votre propos en nous appelant à la prudence et en faisant observer que nous avons révisé les perspectives de croissance deux fois en en l'espace de ces quelques mois. La raison en est très simple, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est que nous sommes arrivés après une motion de censure qui a privé la France de budget. et l'impact de cette motion de censure a coûté 0,2 points de PIB que nous avons retrouvés en passant notre perspective de 1,1 à 0,9. Et puis nous avons eu un événement un peu imprévu dans l'ampleur de ces conséquences, qui est le changement d'administration aux États-Unis, qui s'est traduit par les mesures douanières prises par le président Trump, et nous avons à nouveau pris en compte cela. Et comme je le disais rapidement tout à l'heure, les perspectives de croissance aux États-Unis apparaissent bien à sombrer maintenant, ce qui d'ailleurs d'ailleurs j'espère va pousser l'administration Trump à accélérer ces discussions avec nous. Et nous sommes effectivement dans le déroulé de cette année, dans une situation économique mondiale extrêmement difficile, puisque nous avons ce dialogue qui, j'espère, va s'accélérer avec les États-Unis et l'Amérique. Nous avons par ailleurs une action de la Chine encore plus déterminée, puisque le commerce avec les États-Unis étant largement coupé, ils ont eux aussi un problème d'excédent de production à écouler, raison pour laquelle d'ailleurs avec la ministre nous étions hier à Roissy pour commencer à travailler sur des contre-mesures afin de s'assurer effectivement que l'exécution de ce budget soit respectée en évitant les dérapages, monsieur le rapporteur général, que vous avez signalé. Monsieur le Président, vous êtes revenu aussi sur les incertitudes, sur les risques concernant les recettes, Nous suivons avec la ministre cela mois après mois. Pour le moment, nous sommes au niveau prévu, mais nous resterons attentifs. Madame la rapporteure générale, vous avez aussi rapporté un centre de précision que vous souhaitiez obtenir. Pour une partie, la ministre répondra, pour l'autre, pour ce qui concerne la mise en place de comités de suivi des âgés, qui effectivement résultent d'un amendement. Cet amendement prévoit que cette commission soit mise en place en 2026. poursuivre l'exécution, donc je peux vous confirmer que cette réforme structurelle sera mise en place comme vous l'avez décidé. Je veux revenir sur les propos des sénateurs Grégory Blanc, de la sénatrice Florence Blatresque-Contain notamment, et aussi aux propos du sénateur Stéphane Sautarel. sur le flou, l'incertitude, le refus d'un débat global, le statu quo. Non, rien de tout cela. Rien de tout cela, au contraire. Nous avons prévu, dans un temps beaucoup plus long que celui qui nous a permis d'adopter avec vous et grâce à vous le budget pour 2025, d'avoir une méthode de concertation très large. Cette concertation, elle a été engagée avec la tenue de ce qu'on appelle le conclave sur les sujets de retraite et les travaux se poursuivent. s'engager le 6 mai sous l'autorité de François Repsamène avec évidemment la ministre et moi-même notamment dans le dialogue avec les associations d'élus locaux afin de garantir que les collectivités locales dans leur autonomie contribuent à cet effort de

A ce dialogue, nous allons associer dans les mois qui viennent les élus du Sénat et de l'Assemblée nationale qui le souhaitent, et avec l'ensemble des partis qui souhaiteront y participer, de façon à arriver au mois de juillet à des mesures effectives qui seront celles qui seront issues de ce débat. et je fais appel aux propositions des uns des autres, vous êtes évidemment très bienvenus, et à ce moment-là, le Premier ministre arbitrera, et vous convenez que, pour la préparation d'une loyale finance sur 2026, nous nous y prenons très en amont par rapport à la tradition de notre pays et de nos gouvernements, et ensuite, il n'est pas question que le Parlement soit dépossédé de son autorité, évidemment, mais l'exécutif ayant par le dialogue construit un projet de budget, il sera naturellement présenté aux deux assemblées et nous nous espérons, nous pensons que cette méthode nous permettra d'arriver à une situation qui le fera adopter dans les délais qui vont bien, mais je ne veux pas anticiper, tout cela est très en avant. Alors, revenir sur les commentaires aussi qui ont été faits, notamment, Marc Marc Lamény, vous parlez de Sisyphe, vous vous appelez à des comparaisons internationales. M. Fossin, vous parlez de co-construction, mais je crois que j'en ai dit un mot. Quel est le cadre général dans lequel nous nous situons, précisément au regard des comparaisons internationales et des difficultés qui sont celles de notre pays ? En fait, c'est extrêmement simple. Notre sujet principal, c'est la dette. Ça a été rappelé par la plupart d'entre vous, son 13% du PIB. Le poids de cette dette, 67 milliards, ça dépend des méthodes de comptabilisation cette année, nous allons vers 100 milliards d'euros. L'impératif est de stabiliser les dettes et je réaffirme notre engagement d'être sous les 3% de déficit en 2029. Pourquoi est-ce que cet objectif serait mieux tenu que précédemment ? Parce que si nous ne le tenons pas nous-mêmes, je rappelle que nous sommes sous revue avec perspective négative des trois grands agents de notation. Nous avons des besoins de refinancement importants, et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, ce seront malheureusement des intervenants extérieurs qui vont devoir nous accompagner, ce qu'évidemment en matière de souveraineté, nous ne pouvons envisager. Et pour cela, nous devons protéger la compétitivité. Nous avons un projet qui continue d'être un projet de développement de notre économie. Un projet de développement qui nécessite dans cette concurrence accrue de ne pas augmenter les charges, de ne pas augmenter les impôts qui pèsent sur les Français. Et donc la solution c'est bien la maîtrise de la dépense et c'est bien ce travail que nous suivons sur l'exécution 2025 attentivement avec la ministre et que nous allons engager dans la préparation du budget 2026. Alors, on nous parle à juste titre d'équité et de transformation écologique, mais ça reste évidemment dans ce que nous voulons faire, notamment la transformation écologique. Mais elle demande d'être capable d'investir, elle demande que nos entreprises puissent se transformer. Et c'est donc seulement en ayant cette maîtrise de la dépense publique qu'on pourra financer l'effort à la fois d'équité et de transformation écologique que nous voulons évidemment maintenir. Je veux revenir... Michel Cannevet évoque le courage que cela demande. Ce courage sera un courage collectif, mesdames et messieurs les sénateurs, auquel vous serez naturellement associés, mais sur lequel le gouvernement prendra Alors, M. Maros, j'entends ce que vous dites. Il y a un point sur lequel je me permettrai de revenir sur ce que vous appelez l'activation de la clause de sauvegarde. C'est vrai que l'Union européenne permet d'activer la clause de sauvegarde pour financer l'effort de défense, mais nous n'allons pas activer la clause de sauvegarde, parce que la clause de sauvegarde ce serait de la dette supplémentaire, et des dettes supplémentaires nous n'en voulons pas. Donc c'est à l'intérieur de l'épure que nous vous proposons que nous mettrons en place l'effort nécessaire et éventuellement l'effort supplémentaire de défense. Enfin, Mme Lavarde, vous avez raison. D'abord, merci de souligner l'effort sur les dépenses auxquelles vous avez contribué fortement dans les travaux que nous avons conduits ensemble. Je veux redire que le Parlement continuera d'être associé pour la suite. et je me demandais si je devais revenir après l'intervention de Pierre Barros et la vôtre me conduit à revenir sur le sujet de la retenue à la source, qui m'a valu des courriers fréquents et approfondis avec le rapporteur général du budget. Je ne veux pas être trop long et trop technique, mais puisque vous me sollicitez, J'ai évidemment un respect total pour le texte voté par la Commission mixte paritaire et auquel Jean-François Husson a contribué, dans le cadre aussi d'un avis du Conseil d'État. Et cela étant fait, le gouvernement devait prendre une position en rédigeant un mode d'emploi à destination des opérateurs financiers. Sans entrer dans le détail, dans la décision que nous avons prise, nous avons voulu respecter deux choses. D'abord, la possibilité, même la nécessité absolue pour les services des impôts de pouvoir sanctionner un opérateur qui ferait une opération qui ne serait pas conforme au droit, à l'intérêt général et qui en fait éviterait de façon frauduleuse cette retenue à la source. Et cette possibilité, elle existe, quel que soit le marché sur lequel les acteurs opèrent et dans toutes les circonstances. Et d'ailleurs, ce texte que nous avons rédigé, ne changent en rien les procédures qui sont en cours, d'ailleurs qui se déroulent comme vous savez indépendamment des ministres qui n'interviennent pas. ne reviennent pas, ce qui est d'ailleurs très bien, quand elles se développent. Mais nous avons bien vérifié que ça n'avait pas d'influence sur les procédures en cours. En revanche, l'arbitrage, tel que je le perçois, est le suivant. Les opérations financières peuvent se faire de gré à gré. Dans ces cas-là, on sait forcément quelle est la contrepartie. On peut aller le vérifier. Mais le plus souvent sur les marchés réglementés, elles se font au travers d'une place de marché, de chambre de compensation, qui en fait est la contrepartie des opérations. Et donc, en réalité, si vous vendez un titre sur une place de marché, un titre du CAC 40 sur la place de Paris, et bien, en fait, l'acheteur, c'est la chambre de compensation et vous ne savez pas qui est en face de vous, parce que c'est bien la chambre de compensation qui est en face de vous. Et dans ce cas-là, j'ai pensé qu'il n'était pas raisonnable, si on voulait que les opérations résument, s'il y a Paris, de faire obligation au vendeur ou à l'acheteur de connaître sa contrepartie, parce que la vraie contrepartie, c'est la place de compensation, En revanche, si dissimulé derrière cette place de compensation, il y avait une opération frauduleuse, alors évidemment, qui apparaîtraient, et dans ces cas-là on a besoin de preuves, mais on a vu qu'on les trouvait par des emails, par des SMS entre les opérateurs. Dans ces cas-là, la possibilité de sanctionner une opération frauduleuse et évidemment nous étonnons, parce que je veux procéder à la fois à l'équité et les finances publiques. Pardon de ce développement un peu long, de demander, notamment Mme Lavarde, Mme Lavarde, ne pas devoir me défiler, pardon d'avoir été trop long, et la ministre va compléter mon propos. Merci de votre attention. Merci M. le Ministre, Mme Lenis, je vous donne la parole, je vous en prie. prie. Merci M. le Président. Merci pour ce débat, je dois dire, de très grande qualité, puisque je pense que nous avons beaucoup de choses en partage, même si nous savons que nous avons aussi des différences d'appréciation. Je pense que c'est un très bon signe pour notre capacité à refaire l'exercice du compromis, qui est de facto l'obligation qui est devant nous. Monsieur le rapporteur général, vous avez ouvert ou plutôt conclu votre propos en disant au fond, vous nous appelez à la vigilance et au volontarisme. Et je trouve que c'est précisément, je crois, ce qui nous guide sous l'autorité du Premier ministre ces dernières semaines. Vigilance et volontarisme face aux aléas. Et monsieur le Président, vous avez notamment cité l'aléa notamment sur les recettes d'impôts sur les sociétés. Je voulais vous dire que les 2 milliards de plus sont le fruit des observations comptables de fin d'année et je tiens aussi à vous dire que ces 2 milliards de plus n'ont pas remis en cause notre appréciation de prudence de 1 milliard par rapport à une élasticité mécanique pour que nous ayons dans le cadre total du volume d'IS là quand même de la prudence et donc de la vigilance. Il y a un autre aléa sur lequel vous êtes assez peu revenu ce qui montre que les temps changent mais je veux le citer devant vous qui est l'inflation. Nous sommes face à un scénario d'inflation qui est très difficile à prévoir. Ce matin, nous avions une inflation en rythme annuel sortie à 0,8%, ce qui est faible par rapport encore à des situations que nous avions il y a 18 mois ou 2 ans. Néanmoins, il est difficile aujourd'hui de complètement apprécier la dynamique d'inflation devant nous. D'une part, on a des prix du pétrole qui, vous le savez, sont quand même assez nets recul, ce qui peut être positif au volume de consommation des ménages d'une part, mais qui pèse négativement sur l'inflation, et d'autre part, on a des droits de douane qui, théoriquement, doivent amener à une hausée des prix. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les banques centrales et les meilleurs économistes voient l'inflation comme quelque chose qui est plus difficile à prévoir, et donc je voulais ici le mettre, comme on dit, le verser au compte rendu. Vous avez tous ensuite, vigilance et prudence, rappelé que nous avons effectivement pris un décret d'annulation. Je veux ici vraiment vous rassurer sur le fait que ce ne sont pas des coupes sombres. Nous avons dès le départ, dans la construction du budget, annoncé avec Éric Lombard et sous l'autorité du Premier ministre, que nous avons demandé à l'ensemble des ministères de mettre de côté 0,5% de leur masse salariale et 5,5% de leurs dépenses hors masse salariale. C'est-à-dire qu'ils ne programment pas de les dépenser et que ces dépenses ne puissent être de facto activées que si les temps, la conjoncture, le permettaient. Et c'est ainsi que nous avons créé, dans le cadre de la LoLF, une réserve interministrale de 8,7 milliards. C'est dans ce cadre-là que nous en allumons effectivement 2,7. Et nous avons remis 2,8 milliards de, effectivement, surgel, de dépenses qui n'étaient pas déjà engagées, et qui ont permis de remettre la réserve à 8,7 milliards. Je le dis parce que c'est une pratique qui, je crois, est à la fois respectueuse du Parlement, qui, parce que nous le faisons de manière extrêmement transparente et sincère, et je crois, est une bonne méthode dans un monde avec des aléas. Parce que l'alternative, sinon, c'est de lancer les dépenses et puis, au milieu d'année, de se dire « ah, on arrête tout, je crois que ce serait ni sincère ni respectueux des Français, c'est comme ça que nous procédons ». Ce décret d'annulation, je veux le dire, n'est pas le reflet d'une politique d'austérité générale. sur PIB, 57% de dépenses sur PIB, je ne crois pas que nous puissions parler d'austérité. Vous avez, monsieur le sénateur, dit que vous étiez inquiet des coupsons dans la santé ou l'éducation. Mais reprenons les chiffres de ce que nous avons mis dans le compromis, qui est le budget du pays. Un nom d'âme à 3,4%. Un milliard de plus pour l'hôpital. On ne peut pas parler d'austérité générale. Pour l'éducation, vous savez, des ambitions, vous le voyez d'ailleurs dans les annonces de la ministre de l'Éducation nationale, à la fois de recrutement, de renouvellement de la formation, de recrutement beaucoup plus tôt. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'austérité soit générale. On peut débattre des mesures. On peut dire qu'elles ne sont pas bonnes, si c'est-elle votre avis. Mais budgétairement, je ne veux pas laisser penser qu'un pays qui a 57% de dépenses sur PIB serait un pays dans l'austérité générale. Beaucoup d'entre vous ensuite ont parlé des collectivités et de nos relations entre collectivités et États. Je veux le redire, c'était la réponse d'ailleurs à la question au gouvernement que nous venons d'avoir juste avant. Nous voulons donner de la prévisibilité aux collectivités. Au fond, arrêter cette pièce de théâtre qui commence en général le 1er mardi d'octobre ou sort du chapeau tel un lapin, un chiffre magique auquel tout le monde doit se conformer, qui est source pour les élus qui ont des mandats sur 6 ans pour les maires, parfois 8 ans pour les départements ou les régions en certains cas, totalement ingérable. Et c'est légitime que les collectivités nous demandent d'y voir clair sur là où nous allons. Nous savons où nous allons. Nous allons à 3% de déficit en 2029. De nouveaux maires seront élus l'année prochaine. Il est de notre devoir, de notre responsabilité, de donner au moins la visibilité sur un demi-mandat aux nouveaux élus de 2026. C'est ce que nous allons construire dès la semaine prochaine autour de François Rebsamen. De même, nous devons aux collectivités moins de normes. moins de normes qui entraînent des dépenses contraintes. C'est le rapport de Boris Ravignon, d'Erik Wirth, du Rockler de la simplification qui a été lancé. Je crois que ça va dans le bon sens. Mais là aussi, monsieur le sénateur Sautarel, je ne l'aperçois plus, le mot spoliation ne me semble pas correspondre à la relation qu'il y a entre l'État et les collectivités. Parce que d'abord, je rappelle que les Français n'ont qu'un porte-monnaie. Donc nous ne spolions personne, nous gérons tous avec responsabilité l'argent des français. Point premier. Deuxièmement, la spoliation serait l'incapacité pour les collectivités à amener leur politique publique. Les données que nous présenterons là aussi mardi prochain montrent que l'immense majorité des communes ont des ressources tout à fait stables, que l'immense majorité des régions ont des ressources tout à fait stables, que les EPCI ont des ressources tout à fait stables et que oui, il y a un enjeu, on le sait, sur les départements. Et l'an dernier, La dépense publique en volume augmente 2%, au total. C'est 0,7% de croissance pour l'Etat, 3,1% de croissance pour les collectivités et 3,6% de croissance pour la Sécurité sociale. Il n'y a pas de spoliation. Je le dis ici très fortement parce que sinon on s'éloigne de la réalité. Pour finir, enfin, beaucoup d'entre vous ont parlé des recettes. Et plutôt dans ce côté-ci de l'hémicycle, nous appelons à ce que nous retrouvions des recettes. Nous sommes à 51,3% de PIB, de prélèvements obligatoires et de recettes. 51,3%. C'est un record dans tous les pays comparables aux nôtres. Et je pense qu'il serait fallacieux aujourd'hui 51,3%, il n'y a pas de pays européen au-dessus de nous. Il doit peut-être la Suède et la Finlande. Recette et prélèvement obligatoire, 51,3%. Il serait à mon avis fallacieux de faire croire à nous tous et ici au parlementaire que c'est en augmentant ce ratio que nous allons trouver une solution. Je pense qu'il est utile que nous regardions, et je suis prête à le faire, vous le savez, ce qui mit et ce qui mine l'impôt, les niches fiscales qui ont été très dynamiques dans certains cas, je suis prête à mener le travail, vous le savez, que nous regardions si dans certains cas effectivement nous avons un enjeu d'élasticité à la croissance, très bien, mais créer des nouveaux impôts, augmenter les taux d'impôts, nous pensons honnêtement que la conjoncture ne le permet pas. Les perspectives pour 2026 en un mot. Monsieur Delahaye, vous avez raison. Vous avez raison. Si nous avions et nous voulons vraiment tenir ce principe, si nous avions maintenu nos dépenses de fonctionnement en croissance pas plus haut que la croissance effective de l'économie, nous aurions aujourd'hui un déficit bien plus réduit. Et donc, la perspective pluriannuelle que nous voulons, que les dépenses de fonctionnement n'augmentent pas plus vite que la croissance. Si on avait fait ça, on serait pas à 120 milliards et donc c'est une bonne boussole, je crois, là aussi pragmatique, c'est pas l'austérité. Mais que les dépenses n'augmentent pas plus vite que la croissance, ça paraît un principe sain. Deuxième principe, bien répartir l'effort, madame la rapporteure générale. Vous avez demandé la répartition entre sous-secteurs. de l'effort. Il nous semble que nous ne pouvons pas, et certains d'autres l'ont dit, repartir sur l'idée que l'État porterait près de trois quarts de l'effort de réduction du déficit l'an prochain comme il le fait cette année. C'est trop, c'est pas bien réparti et donc il nous faut mieux répartir entre la sécurité sociale, les collectivités et l'État. Quatrième principe, j'en ai parlé des niches fiscales. Les situations de rente, mille l'impôt. Si nous supprimons beaucoup de niches, eh bien baissons les impôts pour tout le monde. Mais pas que pour quelques ans. Quatrième principe, beaucoup d'entre vous vont nous parler de l'organisation de l'Etat. Le Premier ministre a lancé, comme l'a dit Éric Lombard, et je conclurai là-dessus, une revue méthodique, ministère par ministère, mission par mission. Quelles sont nos priorités ? Comment sommes-nous organisés ? Et notre organisation, c'est non seulement le travail mené par votre commission d'enquête, les agences et les opérateurs qui gèrent de l'argent public au nom des ministères et d'État, c'est aussi la relation État-État déconcentré, à laquelle je sais que vous êtes très attaché pour que ce soit plus efficace et que les préfets et l'organisation territoriale de l'État soient plus au service des politiques publiques, et puis c'est aussi les autorités administratives qui elles sont des régulateurs. C'est très différent de parler de comités en amont de la fabrique de la loi de la norme, de parler d'agence et d'opérateurs qui gèrent de l'argent public ou de parler d'autorité administrative et en plus de parler d'un état déconcentré. Tout ça, il y a des leviers différents. Oui, parfois contribuer à une forme de dépenses publiques, il nous faut tenir. Je tiens à dire qu'agence et opérateurs, il y a deux leviers d'économie. Il y a le levier des dépenses de fonctionnement, d'où les enjeux de fusion, de rapprochement, mais ce sont des économies en quelques milliards d'euros, j'en ai parlé. Mais le plus gros levier, c'est aussi de rapprocher des dépenses d'intervention, que nous y voyons plus clair, que les choses soient pas doublonnées, pas redondantes, pas enchevêtrées. Dernier élément, vous l'avez dit, c'est la méthode. la semaine prochaine la collectivité, au mois de juin la commission des comptes de la sécurité sociale qui sera un moment important, un point d'étape sur cette refondation à l'action publique que le premier ministre veut conduire en juin, en juillet des annonces évidemment sur notre calendrier et nous croyons à la démocratie sociale et je dois vous dire ici mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne lançons pas des ballons d'essai. Ce débat sur les retraités qui nous a beaucoup animé ces derniers jours, c'est simplement le constat que le Premier ministre a confié aux partenaires sociaux une réflexion sur les retraites. Dans le cadre de ce conclave, il et je crois connu, Le 7 mai s'en ouvre un autre à Rome. Je parle de celui qui se tient sous la houlette de M. Maret, qui est laïque et on le sait dédié à l'avenir des retraites. Ce conclave nous dit quoi ? Que le MEDEF, la CPME, le Comité d'orientation des retraites, les syndicats nous disent eux-mêmes que dans la répartition de l'effort entre actifs et retraités, ils discutent d'un certain nombre de mesures dont ce fameux abattement qui a fait la une des journaux. Je le dis ici devant vous, ce n'est pas mon projet de ministre que de le supprimer. En revanche, c'est mon rôle de ministre que de ne pas interdire les débats. Nous leur avons donné carte blanche. Nous leur avons donné carte blanche avec un seul objectif, rétablir l'équilibre d'ici 2030. Il me semble, et je conclurai là, que vigilance et volontarisme pour que nous y arrivions dans un pays fragmenté c'est que nous puissions associer l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des forces vives. Nous n'avons pas le monopole des idées, nous n'avons pas le monopole des solutions. Et donc, par ailleurs, nous devons avoir, à mon avis, une écoute large des propositions. Viendra ensuite la décision. Mais je pense que nous déciderons collectivement beaucoup mieux si nous écoutons tous ceux qui, aujourd'hui, veulent contribuer, comme vous le faites, au rétablissement des comptes publics. Merci beaucoup. Pour la deuxième lecture de la proposition de loi visant à réduire et encadrer les frais bancaires sur succession, la séance est levée.